le procès verbal est donc adopté mes chers collègues par lettre en date du dix octobre la commission des lois demande au sénat en application de l'article cinq de l'ordonnance du dix sept novembre mille neuf au fonctionnement des assemblées parlementaires de lui conférer les prérogatives attribuées aux commission d'enquête pour une durée de six mois afin de mener sa mission d'information sur les émeutes survenues à compter du vingt la conférence des présidents examinera cette demande lors de sa réunion du mardi trente et un octobre prochain l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relative aux services express régionaux métropolitains dans la discussion générale la parole est à monsieur clément beaune ministre chargé des transports

je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour l'examen de cette proposition de loi qui porte un grand projet de transformation de nos mobilités dans tous les territoires de France pour les années à venir. C'est à ce titre, je le sais, un texte attendu par la Chambre des territoires qui, le Sénat tout particulièrement, je tiens ici tout d'abord à remercier l'auteur du texte à l'assemblée nationale le député et présidente de commission, Jean Marc Zoulou de ce sujet majeur il y a quelques mois pour son soutien sans faille ainsi, bien sûr que M. le rapporteur M. le sénateur Philippe Tabar pour le travail très important que vous avez réalisé sur ce texte dans des délais contraints après le dernier scrutin les services express régionaux et métropolitains les Serbes comme on les appellera peut être ont vocation à traduire pleinement l'ambition que porte le gouvernement et je sais grand nombre d'entre vous en faveur de la transformation de nos transports la décarbonation le report modal V. le rail, la priorité au transport du quotidiens qui sont au cœur de notre action et au cœur de cette proposition de loi au fond, il s'agit d'offrir des solutions de décarbonation plutôt que des punitions ou des restrictions. Tous ces éléments se trouvent en effet rassemblés dans le projet de R M tel que nous le concevons et tel qu'il commence déjà à se déployer avec certaines métropoles et régions pionnières. Je pense évidemment à la métropole de et à la région du Grand Est. Pour permettre ce déploiement, nous avons voulu mobiliser deux acteurs reconnus complémentaires, que sont S N C F Réseau et la Société du Grand Paris de les mettre ensemble de manière innovante au service des collectivités et des territoires volontaires comme cela a été envisagé par le Conseil d'orientations des infrastructures, dont jeu saluer encore la qualité du rapport et du travail qui a mobilisé plusieurs d'entre vous comme à l'assemblée nationale, ces deux acteurs ont en effet vocation à travaillerait dans la main pour conduire le dialogue avec les territoires concernés, métropoles et régions, au 1ᵉʳ chef en vue de la réalisation de ces projets nouveaux, c'est ce à quoi nous avons commencé à travailler, c'est ce qui permettra de manière claire, organisée, structurer la proposition de loi qui vous est présentée aujourd'hui. En effet, la question de cette mobilisation commune pour mener à bien ce grand chantier nécessite des adaptations législatives. Celle que propose le texte issu de l'assemblée nationale et déjà amendé par vous, Mᵐᵉˢ et MM. les sénateurs en commission nous semble aller dans le bon sens et je sais que la suite de la discussion parlementaire aboutira à mieux en définir les modalités. Cette mobilisation a vocation à s'inscrire dans un cadre qui définit notamment et c'était attendu, sur le plan politique et juridique l'objet lui même de ces services express régionaux métropolitains

que l'état et des les collectivités doivent mener, conjointement c'est un élément essentiel de notre politique des transports. Ce n'est pas un élément évidemment exclusif c'est important de bien définir l'objet, il est tout aussi important que le cadre que donne cette proposition de loi demeure assez souple, ce soit un cadre de flexibilité d'adaptation au territoire et de confiance dans les collectivités afin qu'ils puissent s'adapter aux réalités forcément spécifique de chacun des territoires concernés. loi de liberté j'espère qu'elle deviendra loi dans quelques semaines est une loi d'adaptation à chaque territoire et je crois que nous devons garder aussi cet état d'esprit, ce sont les collectivités concernées qui devront porter et remonter si je puis le dire des les projets qui seront évidemment au terme de ce texte tel qu'il est aujourd'hui proposé validé par l'état cofinancé par l'état et défini ensuite de manière conjointe et cohérente pour le gouvernement, nous devons prendre pour point de départ les demandes du terrain, c'est l'esprit de ce texte, c'est l'esprit de ce projet, tout entier. Le texte garantit par ailleurs la mise en place de l'ensemble et c'est essentiel des ressources financières nécessaires en matière d'investissements en priorité pour permettre la réalisation de ces services express régionaux métropolitains là aussi, en pleine concertation avec les territoires et en différenciant les solutions d'une métropole ou d'une région à l'autre concernant la question plus largement du financement des Serbes qui, je le sais a soulevé beaucoup de débats au cours des dernières semaines. Parfois, quelques polémiques mais surtout des interrogations je souhaitais apporter d'emblée ici quelques clarifications qui je l'espère pourront vous vous rassurer et nous faire ensemble avancer d'une part l'état a d'ores et déjà prévu des sommes importantes près de huit cents millions de crédits dédiés au service express régionaux métropolitains dans les prochains contrats de plans et de régions qui sont comme vous le savez en discussion région par région c'est une somme qui est très loin d'être négligeable ce n'est pas un premier euro symbolique puisque nous partions dans la génération précédente de zéro c'est un projet nouveau pour lequel l'état mobilise en entrée de négociations une somme déjà extrêmement importante et pour laquelle il est important que les collectivités notamment les régions puissent mobiliser au moins les mêmes sommes c'est une somme qui est consacrée à l'investissement sur une période la période de ces volets mobilités deux mille vingt trois deux mille vingt sept et qui n'ont pas la fin de l'histoire et la totalité de l'histoire du financement des investissements dans les ernest par ailleurs une somme qui a nécessairement un caractère indicatif à ce stade puisque ni le montant exact des projets, ni leur calendrier précis de déploiement ne sont aujourd'hui connus et seront affinés notamment sur la base de ce texte que j'espère devenir loi rapidement pour ensuite préciser les plans d'investissement les plans de financement et les ressources mobilisées pour le dire clairement l'état met une somme importante sur la table il attend que les régions puissent que les régions puissent mobiliser des sommes analogues et bien sûr nous irons ensemble plus loin pour assurer dans la durée le financement de ces investissements est clair qu'entre deux mille vingt trois et deux mille vingt sept pour certains projets en tout cas qui sont aujourd'hui moins avancés que d'autres et qui nécessitent des travaux d'étude ce sont principalement ces études approfondies que nous financeront dans un premier temps et les premiers travaux c'est très important je crois de préciser qu'il ne s'agit donc pas d'un financement exhaustif et définitif de la part de l'état. Je n'ai d'ailleurs par ailleurs, pardon, pas fait mystère de ma volonté de disposer pour les années à venir. Avec vous d'une véritable programmation financière pour les infrastructures de transport, dans lesquelles ces services trouvent naturellement leur place. C'est je crois, d'ailleurs demandé par beaucoup d'entre vous, avec qui j'ai eu, groupe par groupe, la chance d'échanger que je continuerai à Ce que je continuerai pardon à faire dans les prochaines semaines. Le financement des Serbes je le redis doit être partie intégrante de cette visibilité pluriannuelle, quelles qu'en soient les modalités. Il y a donc déjà et il continuera à y avoir des financements et notamment des financements de l'état pour les R M dans leur phase d'investissement en 1ᵉʳ lieu le cas échéant je crois que c'est aussi une des avancées importantes que propose ce texte de loi, des financements innovants tels que des recettes affectées au projet, peuvent et doivent pouvoir être utilisées l'un des actes forts de ce texte est en effet de permettre la création de sociétés de projets, dit le rapporteur, qui pourront, là encore, si les collectivités le souhaitent, au cas par cas, mettre en place une fiscalité locale spécifique adaptée et affectée spécifiquement à ce projet en s'appuyant sur une dette maîtrisée qui, là encore, offre une faculté ne propose pas une obligation mais fait partie de cette boîte à outils du financement des investissements dans les services express régionaux métropolitains est absolument essentiel vous le savez comme je le pense profondément ce modèle a fait ses preuves mutatis mutandis sur le grand paris express et le gouvernement l'a déployé pour les projets de lignes à grande vitesse en cours grâce d'ailleurs à des amendements du sénat dans le p l f pour deux ce mode de financement a plusieurs grands avantages celui d'offrir une grande stabilité du financement une gouvernance spécifique et une mission dédiée notamment une maîtrise d'ouvrage dédié qui sont propices à la bonne réalisation et à l'accélération de ces projets je crois qu'à cet égard l'expertise développée et la mission déployée par la société du grand paris sont exemplaires sais que nous débattrons dans quelques minutes de certains points qui le méritent encore c'est l'intérêt de notre débat de cet après midi le gouvernement notamment est favorable à ce que la priorité du ferroviaire soit clairement affirmée clairement lisible dans la définition de ces services express régionaux métropolitain et que ces services demeurent centrés sur les transports de voyageurs plus que de marchandises ou encore sur la question des tarifs des péages ferroviaires essentiels. Vous connaissez mon engagement à cet égard fassent l'objet d'une réflexion spécifique qui puisse faire l'objet d'un amendement j'espère consensuel ou de compromis que je présenterai dans quelques instants en outre, le Gouvernement a également déposé un amendement pour relever le plafond de dette auquel est soumise la société du grand Paris, ce qui est essentiel par souci de cohérence pour que celle ci puisse remplir ses missions ces discussions pour importantes qu'elles soient ne sauraient remettre en cause le fait que nous nous rejoignons très largement sur les principes sur le contenu sur les modalités retracées dans la proposition de loi telle qu'amendée d'ores et déjà en commission. Je vous remercie très sincèrement pour ce travail rapide, sérieux, engagé dans un esprit constructif constructif par delà les sensibilités politiques. Vous l'aurez compris en un mot le soutien le gouvernement soutient pleinement ce texte. Nous aurons l'occasion de discuter de certains amendements mais son esprit et son contenu sont clairs sa nécessité est avérée et je crois qu'au delà de loi. J'espère qu'elle pourra ainsi

M. le ministre, la parole est maintenant à Philippe Tamaro, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du Développement durable, et ce, pour 10 min. Merci Mᵐᵉ la Présidente, M. le Président le ministre, M. le Président Longo, mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour examiner la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains qui a fait l'objet d'un travail approfondi en commission et ce dans un esprit transpartisane Vous le savez l'objectif est de déployer D R E R métropolitains qui sont depuis lors devenus des Serbes résultent d'une annonce du président de la République en novembre dernier, confirmée quelques mois plus tard par la 1ʳᵉ ministre lors de la présentation du plan avenir pour les transports or vous en rappelez sans doute cette idée n'est pas complètement neuve puisqu'elle trouve son origine dans le rapport annexé à la loi d'orientation des mobilités de deux mille dix neuf c'est didier mandel je me réjouis qu'elle se concrétise aujourd'hui par le biais de cette proposition de loi j'en viens au vif du sujet mais à présent vous exposer les quatre principaux axes qui ont guidé le travail de la commission le premier axe concerne le périmètre des et leurs procédures de mise en place. Notre commission a à cœur de défendre une vision des Serbes décentralisée pensée pour les territoires et adaptés à leur spécificité dans une logique d'équité territoriale. C'est pourquoi la Commission a jugé indispensable d'intégrer systématiquement des lignes de cars express au projet de Ee Mss lignes permettront de relier les métropoles et leurs périphéries les plus éloignées, et ce de manière plus souple et économe qu'à travers le seul mode ferroviaire, les promesses de financement de l'état étant ce qu'elles sont. Il nous revient d'envisager des solutions multimodales qui soient les plus efficientes possible pour nos territoires. Cela est d'autant plus indispensable compte tenu du calendrier très serré prévu par le Gouvernement s'agissant de la mise en œuvre des zones à faibles émissions. Mobilités f e Ce n'est pas notre faute de ne pas avoir alerté à travers un rapport d'information publié en juin dernier en juin dernier sur le risque d'exclure de l'accès aux métropoles. une part importante de nos concitoyens. En outre les infrastructures ferroviaires modernisées ou même construites dans le cadre seront pas disponibles du jour au lendemain. Il faut donc que chacun puisse bénéficier au plus vite de moyens de transport collectifs adaptés c'est également la raison pour laquelle la Commission a adopté un amendement précisant que la décision de mettre en œuvre le contrôle et les sanctions du respect des règles applicables à la f e tient compte le cas échéant, de l'avancement des Serbes Cette mise en cohérence est à mes yeux essentielle

Pas d', copartageants, c'est un peu de l'écope également. J'en viens à mon 2ᵉ axe, qui est un sujet de préoccupation majeur de notre Commission. Il est essentiel que la procédure de création des S serbes prennent de racines dans les territoires et notamment dans les régions. Dans cette perspective, la Commission a confié au Conseil régional chef de file des mobilités le soin de proposer par une délibération la création d'un Er M. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille écarter les autres collectivités territoriales du processus. Les Serbes nee peuvent fonctionner que sur la base d'une volonté territoriale et d'objectifs définis et partagés entre tous les acteurs locaux, notamment les départements et les mers. La Commission s'est également penchée sur les enjeux de gouvernance en veillant à son caractère collégial transparent et tourné v.. La qualité de service et et la sécurité des Serbes à ce titre, la Commission s'est aussi montrée particulièrement vigilante aux conditions d'intervention de la Société du Grand Paris, rebaptisée Société des grands projets. Nous avons souhaité renforcer le rôle des collectivités dans le choix de la Gp comme maître d'ouvrage, et ce n'est donc qu'à la demande de la région et des autorités organisatrices de la mobilité concernée de la mobilité Sous réserve ensuite d'un accord du ministre chargé des transports, puisqu'il est question du réseau ferré national propriété de l'état, M. le Ministre, il n'en va pas de même des lignes ferroviaires transférées en gestion ou en propriété aux collectivités territoriales pour lesquelles la Commission a garanti la possibilité de choisir ou non de faire intervenir l'g P en tant que maître d'ouvrage. 3ᵉ axe, c'est dans le prolongement de ces questions la Commission s'est montrée attentive à garantir la bonne articulation des interventions de la G P. D'une part, de la N C F Réseau et de sa filiale Gare Connexion, Connexion, d'autre part, qui assurent respectivement une la gestion du réseau ferré national et des gares de voyageurs. À ce titre, la Commission a confirmé le principe de répartition des responsabilités proposé par l'assemblée nationale la P pourra ainsi intervenir en tant que maître d'ouvrage essentiellement sur des infrastructures nouvelles. du réseau ferré national mais aussi pour des infrastructures non utilisées depuis cinq ans ainsi que pour des projets d'infrastructures de transport public, urbain ou périurbains, en correspondance avec l'une des gares ferroviaires d'un cerf. Ainsi, la G P pourra apporter au déploiement des futurs Serbes toute l'expérience acquise dans le cadre de la réalisation du Grand Paris Express. Je rappelle et nos collègues franciliens le savent très bien qu'il s'agit nii plus ni moins du plus grand projet d'infrastructure d'europe. Elle pourra également faire bénéficier les projets de Serm de sa capacité d'emprunt, ce qui est un atout non négligeable, pour autant, il n'est pas évident évidemment, question d'archipels le réseau ferré national, qui relèvera toujours de S N C F. eaux. La Commission a donc été très attentive à clarifier encore davantage le périmètre et les modalités d'intervention de la G P dans le cadre des Er Ps, de même que les conditions de remise des ouvrages aux futurs gestionnaires d'infrastructures. Quatrièmement, j'en viens à ce dernier axe qui est relatif au modèle économique et financier des Serbes des Serbes qui reste pour l'heure la grande la grande inconnue malgré vos proposs rassurants M., le ministre, en effet, ce texte ne règle en rien la question du financement des services express régionaux métropolitains que ce soit en investissement ou en fonctionnement or alors que leur déploiement suppose des dizaines de milliards d'investissements tant en matière d'infrastructures que de matériel roulant ferroviaire l'engagement de l'état est à ce jour très loin d'être à la hauteur une enveloppe d'un montant de seulement sept cents millions d'euros mais plutôt huit cents millions d'euros si j'ai bien entendu parce que c'est sept cents que le président de la république avait annoncé alors même qu'il y avait huit cents millions d'euros que vous aviez promis avant l'été mais vous nous avez confirmé qu'on était plus sur huit millions pour financer au mieux c certaines études préalables au delà des besoins d'investissement se poserait inévitablement la question du financement de l'exploitation des serbes de l'expérience du grand paris express est à cet égard éclairante et malheureusement inquiétante je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en discuter lors du prochain du projet de loi de finances pour deux mille vingt quatre de même que s'agissant des effectifs de la g p qui voient le champ de ses missions élargi par la présente proposition de loi sans que ses moyens humains ne soient renforcés pour autant avant même de cette échéance la commission a adopté le principe de l'organisation d'une conférence nationale de financement des er ms d'ici le trente juin deux mille vingt quatre cette réflexion collective nee préjugera pas des modalités de financement qui seront retenues in fine dans chaque territoire en complément chers collègues et afin d'éviter que le déploiement des serbes se traduise par de moindres investissements dans la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire la commission a prévu ferroviaire, la conclus par l'état et la n c f réseau on ne reviendra pas sur ce contrat, on a dit beaucoup de choses le programme annuel des investissements de cette dernière en faveur du réseau. Enfin, avant de conclure, je vous indique que je vous soumettrai tout à l'heure un amendement visant à garantir la sécurité des usagers des futurs Serbes à travers la conclusion systématique d'un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports. Je ne serai pas plus long je vous remercie de votre attention

madame la présidente monsieur le ministre monsieur le rapporteur chers collègues c'est en novembre dernier qu'emmanuel à la surprise générale sa volonté de développer le service ferroviaire dans treize métropoles françaises pour un coût de sept cents millions d'euros s'en est suivie tout un tas d'annonces pour le secteur du ferroviaire où en avril où en avril elisabeth borne première ministre annonce un plan de cent cent milliards d'euros dans le cadre d'un plan de développement puis la tournée des médias du ministre délégué chargé des transports quii évoque des pistes de financement pistes de financement comme la taxation des sociétés d'autoroutes et donc indirectement des usagers de ces autoroutes privatisées ou encore la taxation du secteur arien. En réalité ce plan de 100 milliards n'est pas ficelé Personne ne sait quand les Serbes seront opérationnels ni qui les financera. Enfin, si il existe une grande probabilité que ce soit les Français les pluss modestes, qui sont encore mis à contribution pour un gain d'efficacité quasi inexistant dans les zones rurales. La proposition de loi place le ferroviaire comme élément indispensable de la construction des métropoles, avant même la vision des mobilités à long terme pour l'ensemble des Français. des Français. la mise en place, encore une fois, de financement à hauteur de plusieurs milliards d'euros dans les zones urbaines, sans le moindre bénéfice pour les Français des zones rurales. Chers collègues, ce texte risque d'aggraver les fractures qui existent au niveau national entre les zones rurales et les zones urbaines et périurbaines. L'article un est en ce sens assez clair, étant à réserver le stationnement dans les gares, épaules pôle d'échange aux vélos, véhicules de covoiturage et autres moyens de mobilité partagés cela signifie qu'un habitant en zone rurale ou périurbaines. seul mais prêt à consentir de faire l'effort de laisser sa voiture pour se rendre en ville en train est exclu des gares et pôle d'échange Pire il nee pourra pas non plus se rendre en ville avec sa voiture, puisque vous refusez de suspendre les zones à faible émission mobilité. Les pluss riches seront libres de se mouvoir et les plus pauvres cantonnés chez eux. nous avons besoin de garanties sur le fait que les zones rurales seront dés enclavées, que les habitants des zones ne seront pas encore une fois les grands oubliés La France a besoin d'une loi de programmation des transports et pas de textes saucissonnée par ci par là, en empêchant toute vision à long terme. De nombreux projets doivent être étudiés et la qualité du réseau routier, notamment des routes secondaires doit aussi devenir une priorité mais au fond M.. le Ministre, tout ce projet, ce refus de favoriser la mobilité des Français habitant en zone rurale nee sert souvent qu'axées qu'aux électeurs ce qui se trouve essentiellement dans les grandes villes, est à proximité en punissant d'une certaine façon ceux qui, selon vous, votre malade.

Mᵐᵉ la Présidente, M. le Ministre, mes cher chers collègues, dans le cadre des objectifs que la France s'est fixés en matière de transition écologique, les services express régionaux métropolitains par la présente proposition de loi constituent une innovation structurante pour nos territoires, je souhaite saluer le travail consensuel effectué par notre rapporteur Philippe Tabar, la commission Tamaro, la commission de l'aménagement du territoire du développement durable et le gouvernement il est vrai que pour être acceptés par tous les projets liés à la transition écologique méritent un travail concerté et approfondi allant dans le sens de l'intrat des franais surtout lorsque cela concerne les mobilités s'agissant des investissements liés à la réalisation des services express régionaux métropolitains une unanimité se dégage les besoins de financement sont extrêmement importants dans l'immédiat ils ne sont pas au rendez vous les sept cents millions d'euros annoncés par emmanuel macron sont dérisoires au regard du coût du déploiement des di serm d'ici dix ans estimé a minima autour de quinze milliards d'euros infrastructures de transport et matériel roulant compris au moment de déterminer leur position sur ce texte les sénateurs du groupe Les indépendants ont particulièrement insisté sur ce point notre groupe n'a de cesse de rappeler que la transition écologique a un prix. C'est pourquoi nous saluons la création de la conférence nationale de financement, qui aura pour mission de dégager des solutions pérennes en la matière. L'état ne pouvant pas tout à l'évidence, il nous faudra trouver des financements publics, certes, mais aussi à aller chercher des solutions avec le secteur privé. Si les moyens financiers constituent le nerf de la guerre pour le déploiement des ermes. Il nous faudra lever d'autres incertitudes principalement techniques, plusieurs sénateurs ont soulevé des impossibilités de nature opérationnelle. En effet, dans de nombreux territoires, je pense à l'hérault ou à la Loire Les sillons ferroviaires sont déjà au maximum de leur capacité. Le but n'est certainement pas de mettre en place des termes en Eure creuses nos citoyens ont de réels besoins de mobilité. C'est pourquoi je me félicite que la réflexion nee se limite pas aux étoiles ferroviaires et que l'intermodalité soit fortement encouragées. cette complémentarité est fondamentale

me réjouis donc de voir jeter les bases d'une coopération entre la s n c f réseau et la g p nous serons attentifs à ce que cela produise des bénéfices avérés pour les usagers et les territoires. Je tiens, à ce sujet, à mettre l'accent sur la place des collectivités territoriales, régions et départements surtout, qui a été dégagée par la propositionnel poursuivre sa marche décentralisation décentralisation Cctv à la manœuvre sur ces questions de transport collectif marque sans aucun doute une 1ʳᵉ étape du renouveau démocratique que représente la décentralisation des décisions. nous pouvons nous en féliciter faisons confiance à nos parfaitement leurs besoins et particulièrement à nos mères les consulter en amont du déploiement d'un projet de service express régional métropolitain sur leur territoire, relèvent de l'évidence le rôle l'évidence le rôle des maires au plus près de nos concitoyens et des usagers permet de faire émerger des solutions équilibrées et réalistes. mettre les acteurs concernés autour de la table au delà du respect dû aux territoires et à leurs spécificités. C'est assurer une réponse en harmonie avec la nécessité des bassins de vie que serviront les R E R métropolitains même si le chemin reste long. Les projets de serme semblent avec cette proposition de loi pouvant être lancés sous les meilleurs auspices. Le groupe les indépendants restera toutefois vigilant sur les questions relatives aux moyens financiers et techniques pour lesquelles les solutions pérennes n'ont pas encore été trouvées. Il votera en faveur de ce texte afin d'accélérer et de consolider ce processus supplémentaire de transition juste pour nos territoires. Chers collègues, la parole est maintenant à M. Franck Decin, pour le groupe Uno, centriste, pour une durée de 8 min.

Mᵐᵉ la Présidente, M. le Ministre, chers collègues, j'ai l'honneur de m'adresser à vous depuis cette tribune pour la 1ʳᵉ fois. Je suis particulièrement heureux que cette 1ʳᵉ intervention en tant qu'orateur de mon groupe Union centriste, puisse porter sur les R R métropolitains, R métropolitains, dont je connais à la fois l'impérieuse nécessité, mais aussi

La présence de moyens de transport modernes fiable et décarboné ne peut demeurer le seul apanage de la région capitale. Le temps est venu d'équiper nos grandes métropoles de réseaux de transports à la hauteur de leur poids économique et social. Alors que la livraison des 1ᵉʳˢ ouvrages construits par la G P pointe son nez avec le prolongement au nord et au sud de la ligne quatorze métro parisien faisant d'elle un mondial d'efficacité et de modernité je crois qu'il faut saluer mais surtout se rendre compte du travail effectué par la société du grand paris depuis sa création en en seulement treize années cette structure passée de quelques dizaines à mille collaborateurs environ est en train de mener à bien le plus grand chantier d'europe cela a été dit par l'ensemble des orateurs il s'agit ni plus ni moins de doubler en moins de vingt ans la taille du réseau de métros parisiens existants, ce qui est absolument colossal Le grand Paris Express a nécessité la création de cette société ad hoc qui n'avait jusqu'à maintenant vocation à perdurer dans le temps ces dernières années. Il est apparu qu'il serait malheureux pour ne pas dire regrettable de se passer de cette expertise accumulée au cours des années dans cet esprit ce texte, fruit d'un travail de concertation entre la S N C F réseau et la G P porte des mesures de coordination de simplification, qui permettront de décliner au local des solutions de transport ambitieuses en respectant les souhaits des collectivités au sein de structures juridiques dirigées par Pour Pour que les termes soient un succès, il faudra que la société des grands projets, les collectivités ainsi que N C F, réseaux et Gare et connexions mettent en place, dans chacun de ses projets locaux, un dialogue franc sincère. apaisé. le compromis trouvé à l'occasion de ce texte me laisse penser que chacun de ces acteurs est prêt à afin de parvenir au meilleur résultat en termes d'efficacité et surtout de rapidité. Je souhaiterais néanmoins appeler votre attention, chers collègues, sur deux points particuliers dont, je l'avoue, j'ai du mal à saisir la pertinence Dans nos régions respectives, nous connaissons des exemples où la mise en place d'un serre nécessitera des travaux importants sur de l'infrastructure exploitée que ce soit une voie circulée ou une gare de voyageurs prenons l'exemple de la gare de Marseille Saint Charles. Hein, il est évident que la mise en place du serme d'aix Marseille nécessitera une refonte intégrale de la gare Saint Charles, avec une mise en souterrain d'une partie importante des circulations telle que la proposition de loi est écrite aujourd'hui l G P nee pourrait pas intervenir sur un tel chantier car cette gare car cette gare est en exploitation, souhaite souligner le caractère un peu illogique de cette rédaction. Pour tirer bénéfice à plein d'expertise accumulée il faut permettre au ministre, à vous, M. le ministre des transports, et aussi aux collectivités concernées, de décider au cas par cas e des solutions de maîtrise d'ouvrage les plus appropriées.

Je crois que cette doit être facilitatrice et non restrictive, il me semble qu'il serait bon aloi de laisser au pouvoir réglementaire ainsi qu'aux collectivités les possibilités de décider, pour eux mêmes, au eux mêmes, au local, des solutions les plus adaptées à leur territoire. Même si le financement des Serbes n'est pas l'objet de cette P l je crois que nous avons je crois que nous avons un devoir de vigilance sur ce point cela a été aussi rappelé par les orateurs il ne faut pas promettre des miracles sans pouvoir les financer

quii est nettement insuffisant enfin vous avez qualifié vous tout à l'heure dans votre discours de somme à caractère indicatif donc je suppose que Ça ne peut être que plus dans l'avenir, donc la question du financement des investissements lourds. Absolument entière. Je crois que, là encore, le modèle du Grand Paris Express doit constituer un exemple à reproduire le financement de l'investissement doit être pensé dès le début de la phase de conception afin de permettre à l'ensemble des acteurs d'avoir une vision claire des tenants et aboutissants du projet quand il est question d'infrastructures à plusieurs milliards d'euros et de plans de financement pluriannuel enjambant dans de nombreux cas les échéances politiques locales, ces derniers doivent être limpides et anticipés, Il nous faudra faire preuve de créativité dans les ressources financières à mobiliser le modèle de fiscalité affecté propre au grand Paris Express ne pourra pas être reproduit à l'identique dans noss différentes régions, à l'évidence l'assiette fiscale Yy est plus faible et nee permettra pas de lever des sommes sur les marchés à des taux aussi compétitifs Je doute et et je ne suis absolument pas favorable, vous le savez, à, à une fiscalité locale supplémentaires et à des impôts locaux supplémentaires pour nos territoires. J'appelle donc solennellement l'état à prendre sa part dans le financement de ses infrastructures. a minima il faudra qu'un débat s'engage dans les prochains mois sur les modalités de financement de ces termes qui demeurent pour l'instant tout à fait je dirais obscur je salue à cet égard, euhh l'amendement. Ce rapporteur de la Commission visant à la sécurité à sécuriser la tenue d'une conférence de financement des Ser Ms, ce sera un un moment très important, un rendez vous très important. De manière analogue, à plus long terme, il nous faudra également lancer une refonte du financement de l'exploitation de ces infrastructures, ce qui nécessitera une discussion franche sur la manière de donner aux collectivités les moyens nécessaires au bon fonctionnement de nos transports publics. Il nous faut, à tout prix, éviter nous avons connus récemment afin d'aider nos collectivités à s'engager dans ce magnifique projet national que peut constituer la création de ces termes aux quatre coins de l'hexagone. Mon groupe votera donc sans aucune réserve en faveur de ce texte. Je vous remercie.

d'offres de service, des transports du quotidien pour au moins au moins une grosse dizaine de nos métropoles, notre pays accuse un net retard, nombre de nos projets n'avancent pas juste ceux du léman express de strasbourg et de bordeaux ont d'ores et déjà atteint des niveaux significatifs l'ambition c'est tout simplement d'en finir avec cette lourde réalité qui fait que quatre vingt dix des déplacements entre dix et quatre vingts kilomètres se font en voiture et la plupart du temps seuls dans sa voiture en grande périphérie des villes la part modale des transports collectifs chute brutalement par rapport aux agglomérations centre on passe de vingt sept dans les pôles à cinq dans les couronnes c'est donc là que réside le potentiel le plus important de décarbonation compte tenu des longues distances quotidiennes parcourues en véhicules individuels c'est toute l'ambition des fermes celle de la cohésion territoriale de la république face qui peut déterminer une trajectoire financière mais

personne nee peut nier la nécessité de construire des trajectoires financières pour assurer les coûts d'exploitation des fortes augmentations de services et des investissements nouveaux parfois nécessaires en ce sens Nous saluons l'apport du rapporteur proposant des tarifs de péage ferroviaire plus supportables dans les périmètres des Serm, l'apport aussi d'une conférence nationale de financement des ermes les amendements socialistes pour la construction de trajectoires de financement. Le texte identifie les éléments d'une labellisation Le rapporteur a eu raison de rehausser l'importance des cars express. de la même façon. L'intégration à part entière des réseaux cyclables sera un formidable accélérateur d'intermodalité et de décarbonation. texte propose des dispositions pour faciliter une gouvernance pas évidente entre régions

qui ont besoin de mobilités quotidiennes, fluides et pratiques et qui se contrefiche, Passez moi l'expression des prés carrés de nos différentes collectivités nous ne pouvons donc pas au Sénat supprimer, abruptement de ce texte la nécessité d'aller V.. une bii éthique intégrée bien sûr le mieux est souvent l'ennemi du bien l'amendement de rétablissement que nous proposons a le souci de la nuance de la nuance pragmatique qui pourrait être un compromission ne réduisons pas le rôle de l'autorité organisatrice des mobilités porteuses d'un projet Serm E M et l'importance de la dynamique qu'elle pilotera elle n'a pas besoin que la loi lui impose de consulter chacun des maires elle le fera naturellement sa délibération est importante comme celle de la région pour demander à l'état la reconnaissance du statut de E M au projet Mon groupe propose des amendements là dessus La nouveauté déterminante c'est la vocation c'est la vocation nouvelle que ce encadre pour la société du grand Paris partant du constat des acquis de cet établissement public il serait dommage en effet de démanteler tout cela après le Grand Grand Paris Express réalisé la société des grands projets, c'est la possibilité de conditions d'emprunt favorables. pas de carcan d'annualité budgétaire, la faculté de taxe affectée locale et, bien sûr, l'expérience et l'expertise de ces équipes. Il était essentiel de garantir l'unicité de la gestion du réseau ferroviaire, Notre rapporteure a amendé pour préciser que c'est à titre gratuit que réseaux et gares et connexions récupéreront les infrasons il serait incompréhensible M.. le ministre que le gouvernement et l'assemblée nationale veuillent supprimer cette précision essentielle. Deux dispositions ajoutées en commission sont à notre sens contreproductives et il faudrait y revenir aujourd'hui vouloir conditionner mécaniquement les contrôles et les sanctions des f eu à l'existence d'un serme avancé à l'apparence d'une bonne idée se seraient inévitablement utilisé comme un prétexte à l'immobilise dans la lutte contre la pollution de l'air d'origine automobile ce serait aussi je le crois bien une petite entorse à l'article quarante cinq et au périmètre de cette p p l p l il serait de même singulier de détourner l'esprit du zan zéro artificialisés nette en imputant imputant la consommation foncière occasionnée par les r m au forfait national, alors que ce sont des projets d'intérêt régional dans le cadre du forfait régional. on sera sans doute plus attentif à la consommation d'espace pour conclure cette proposition de loi est positive. Ces dispositions seront utiles pour faciliter la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains, leur donner de la cohérence, de la pour provoquer aussi une clarification et une sécurisation des financements nécessaires. mon groupe la votera. Merci beaucoup, chers collègues, la parole est maintenant à M. Pierre Barros, du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste kanakis pour une durée de 5 min.

madame la présidente monsieur le ministre monsieur le rapporteur chers collègues nous passons beaucoup de temps dans les transports notamment en voiture à elle seule elle représente soixante douze

on est attaché à la bagnole on aime je l'adore, déclarait récemment le président de la République, c'est sans doute ce qui explique son peu d'ambition pour le ferroviaire et pour les alternatives à la voiture au camion héritier des politiques d'aménagement du territoire qui sévissent depuis les années 60 et favorisent le tout automobile. Les Français aimeraient pourtant pouvoir se déplacer facilement sans que cela leur coûte trop cher s'ils prennent malheureusement leur voiture, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. La mobilité est un droit qu'il nous faut réaffirmer en octroyant de réels moyens au transport collectif et aux services publics, il faut les rendre davantage accessibles et efficaces pour développer la qualité de vie et lutter contre le dérèglement climatique nous discutons aujourd'hui d'un texte qui est passé par le filtre de l'assemblée nationale puis par celui de la commission d'aménagement du territoire et du développement durable J'aimerais saluer les travaux qui ont été réalisés collectivement par la Commission et qui améliorent nettement la version initiale à travers cette nouvelle proposition de loi, j'entrevois une volonté claire de matérialiser un véritable maillage de transport dans les grandes agglomérations du pays. L'intermodalité s'inscrit au cœur des services express régionaux métropolitains grâce au projet de déploiement de R. E. R. métropolitains. Sincèrement qu'ils aboutiront, tout cela reste tout de même du domaine de l'hypothèse, car si nous saluons les intentions il reste à déterminer les moyens notamment financiers qui seront mis sur la table j'ai bien noté monsieur le ministre les moyens conséquents qui sont mis et évoluer la les enveloppes mais ça reste à confirmer malgré tout le président de la république annonçait fièrement fin septembre qu'il y aurait sept cent maintenant huit cents millions d'euros dédiés au erreur métropolitain j'ai bien compris aussi que c'était pour commencer les études mais c'est un chiffre très important certes mais tous les travaux du sénat annoncent plutôt un effort minimal entre quinze et vingt milliards d'euros pour développer les lignes imagines par le d'orientation des infrastructures ces huit cents millions paraissent donc bien dérisoires et nous serons très attentifs lors du projet de loi de finances deux mille vingt quatre à défendre les moyens nécessaires au développement des transports ferroviaires

c'est une très grande et bonne idée mais il faudra aussi apprendre des erreurs, notamment celle du Grand Paris Express, qui n'a pas su tenir les coûts, le calendrier et qui aura contribué à artificialité ou rendre inexploitable nombre d'espaces agricoles en île de France. Monrose proposa tout de même de limiter le recours à des prestataires externes. Tant nous devrons profiter des atouts et des compétences des acteurs publics plus à même de porter l'intérêt général qui nous tient à cœur ainsi vous l'aurez compris nous trouvons ce texte porte des intentions claires pour décarboner les mobilités mais que des améliorations sont possibles. Nous vous les soumettrons en séance pour pouvoir aboutir à un texte auquel nous serions davantage favorables. Donnons nous des objectifs de report modal réellement efficaces, garantissons des financements de la part de l'état, soyons exigeants sur la qualité des aménagements, des pôles d'échange multimodaux, sur la qualité des services proposés et des fondons un prix du billet supportable pour les usagers c'est le sens à donner à ces nouveaux services express régionaux métropolitains dans le cas contraire les bases que nous posons avec ce texte seraient de n'être qu'un affichage de plus, offrant simplement un label qui ne répondra ni aux besoins des usagers, ni à nos territoires, ni à l'urgence climatique. Merci beaucoup, chers collègues, la parole est maintenant à Mme Véronique Ge Guillotin, du groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 5 min.

des discussions générales de mobilité, que la raison grand test est fort impactée par ce par ce texte c'est avec un grand plaisir que je me présente aujourd'hui quatre ans qui ont été nécessaires depuis les priorités dessinées dans la loi d'orientation des mobilités de deux mille dix neuf pour enfin développer un cadre légal permettant d'accélérer le développement des mobilités du quotidien tout en désenclavement nos territoires et en offrant à nos concitoyens de nouvelles offres de mobilité adaptées et décarbonées le groupe d s e qui partage le souci de l'équilibre entre les territoires souscrit naturellement aux objectifs et ambitions de cette proposition de loi. Les enjeux de développement de nos territoires sont plus que jamais cruciaux pour l'équilibre de notre pays où la fracture sociale et économique s'intensifie face à la métropolisation de notre développement économique, tirée par une tendance à la concentration géographique des emplois cadres, il faut effectivement la capacité à nos périphériques de faire réseau avec leurs pôles d'attraction devant ces défis multiples et transversaux. Nos réponses doivent impliquer tous les acteurs concernés en ce sens. Nous félicitons les travaux qui ont été menés par le Sénat lors de l'examen du texte en commission et notamment par son rapporteur, Philippe Tamaro. Les services express régionaux métropolitains doivent être pensés par et pour les territoires et c'est bien l'esprit de la Commission. Les collectivités territoriales, désormais placées au cœur du processus de décision, se sont enfin vu attribuer les outils de coordination nécessaires Cependant, au delà d'être collective, notre réflexion devra d'emblée être multimodale plus que de simples Ee R métropolitain les services expression aux métropolitains seront de véritables choc d'offre pour les transports collectifs. Les cernes doivent pouvoir tirer le maximum de la complémentarité entre les transports collectifs routiers et ferroviaires afin de répondre au mieux à l'urgence climatique aux inégalités et particularités territoriales ainsi qu'aux aspirations des Français en matière de mobilité dans leur bassin de vie une offre de cars à haut niveau de services le développement de réseaux cyclables et la promotion du covoiturage et de l'autopartage devront systématiquement accompagner le déploiement des Ser Faciles à mettre en place et peu coûteux, ils permettront de répondre à l'urgence impérative de décarbonation des mobilités et d'accompagner la mise en place des F e en évitant d'exclure certains usagers du cœur des villes, une préoccupation dont ma collègue, Nathalie Delatte sest attachée à travers l'adoption en commission de son amendement visant à ce que la mise en œuvre des dispositifs de contrôle et de sanctions du respect des règles D F F tiennent compte du déploiement des Er notre groupe est profondément convaincu que z f i sem sont complémentaires qu'il ne faut pas les opposer afin d'atteindre nos obligations écologiques et améliorer la qualité de l'air et de vie des Français à conditions de répondre aux exigences d'acceptabilité et de justice sociale, Or, nous ne pouvons pas pénaliser nos concitoyens qui recourent à la voiture individuelle, s'ils n'ont pas encore d'alternative crédible et efficace Néanmoins, Si partager les objectifs de ce texte est une chose. Nous ne pouvons faire l'impasse comme les groupes l'ont fait précédemment sur les financements Je ne vous apprends rien. Si je vous dis que l'argent est le nègre et que dire choc d'offres d'offre de services quelquefois veut également dire mur de financement cette proposition de loi nee fixe en effet pas les garanties de financement et ce n'est pas son objet ce qui constitue quand même un motif d'inquiétude à ce jour l'état annonce un déblocage et vous l'avez dit monsieur le ministre de huit cents millions d'euros en faveur des ser ms mais on sait que la note se comptera en plusieurs dizaines de milliards d'euros avec différents projets de différentes natures et auteurs de financement le plan de nouvelles donnes ferroviaires de l'ordre de cent milliards d'euros d'ici deux mille quarante nee précise pas encore le les montant attribué au développement des serres nous serons donc extrêmement attentifs et vigilants aux réponses qu'apportera la conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains organisée d'ici le trente juin par ailleurs passer l'investissement dans l'infrastructure c'est toute une qualité d'exploitation qu'il faudra assurer du matériel roulant aux gares en passant par le personnel et la programmation des sillons et des expériences, notamment à Strasbourg doivent attirer notre groupe déposera un amendement en séance afin d'éclaircir le du périmètre d'établissement des fermes, aucun territoire, aucune commune soumise à Aertec ne doit être oubliée que ce soit dans le processus de concertation initiale ou dans le déploiement effectif du de Il nous semble en effet nécessaire d'établir un périmètre précis, objectif permettant d'éviter une aspiration des financements parés pour les métropoles, auquel cas la cible principale du texte serait manquer, à savoir le désenclavement des territoires ruraux et périurbains, l'enjeu de ce texte n'est pas celui de la mobilité il s'agit effectivement de construire ensemble l'aménagement durable des territoires où liberté d'action flexibilité souplesse opérationnelle, devront être ces nouveaux dogmes. Naturellement, le groupe D S E votera favorablement cette proposition de loi. Merci, chers collègues, la parole est maintenant à Mme Nadège Nadège Avez du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendant pour une durée de 7 min. Merci, Mᵐᵉ la Présidente, et je profite de cette prise de parole pour vous féliciter de votre élection à ce poste, M. le rapporteur, M. le Président de la Commission, M. le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi dont nous partageons l'esprit sur tous nos bancs,

qui s'appuie sur l'ossature existante et la réouverture de lignes oubliées, Il nous faut pour ce faire, non seulement augmenter la fréquence de passage et les amplitudes horaires, mais aussi bien entendu, mieux irriguer les alentours des grandes villes concernées afin de désenclaver les territoires insuffisamment connectés périurbains et ruraux. Sur le modèle des Ee r franciliens, mais avec l'impératif de déclinaisons propre à chaque réalité territoriale et j'y reviendrai il est aussi question évidemment de répondre à l'urgence environnementale avec une accélération de la planification écologique rendue possible par de nouvelles offres de mobilité adaptée et décarbonée. La 1ʳᵉ ministre le soulignait en février, c'est lorsque nos concitoyens pourront trouver un transport en commun régulier, facilement accessibles et fiables qu'ils pourront réduire leur usage à la voiture. Le groupe D P I soutient pleinement l'ambition et le dispositif porté par ce texte déposé par le député Jean Marc Zuléma à son action adoptée en 1ʳᵉ lecture à l'assemblée nationale avant l'été. Notre commission l'a approuvé mercredi dernier et je salue notre rapporteur, Philippe Tabar pour son travail. Cette avancée législative s'inscrit en continuité d'engagement déjà pris, notamment dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités faisant suite à cette promulgation et au rapport du conseil d'orientation des infrastructures en deux c f réseau avait alors élaboré un schéma directeur dans le but de désaturer les étoiles ferroviaires et de développer ses services express cette nécessité d'une meilleure desserte a été défendue par le Président de la République en novembre dernier. Il l'a réaffirmé, en septembre, à l'issue du conseil de planification écologique, une priorité nationale qui trouve ici une déclinaison attendue dans le dispositif des termes qui entendent transformer la mobilité pour des millions d'usagers l'inter et la multimodalité tiennent une place fondamentale s'il est évidemment question d'infrastructures. L'ambition s'inscrit dans un aménagement bien plus global de notre territoire, d'une réflexion approfondie dès la conception non seulement sur l'intégration des services existants, mais aussi sur une offre élargie, pas d'opposition mais une complémentarité entre les déplacements en commission, les réseaux cyclables et les lignes de transport routier à haut niveau de service ont été incluses dans la définition des termes, de même que le cas échéant le covoiturage et l'autopartage en plus du transport fluvial, la création et l'adaptation de gares

j'y faisais référence, il existera autant de Serbes que de territoire retenus en outre, afin de confirmer le rôle de chef de file des mobilités de l'échelon régional. La Commission a prévu qu'une délibération du Conseil régional concerné soit prise pour décider de créer une M. nous y sommes là encore favorables. Nous soutenons également le principe d'un renforcement de la collégialité entre les maîtres d'ouvrage et de l'implication des financeurs, Autre objectif faire intervenir un maître d'ouvrage dans ce déplacement la S G P, dont l'expertise reconnue, ne doit pas être perdue mais partagée il s'agit de décliner un modèle à la française, reconnu à l'international, disposant d'une importante capacité d'emprunt et d'un fonctionnement souple mais il ne s'agit ni de centraliser la gouvernance des R M, ni d'en faire un concurrent avec la N C F. F. G P devra permettre la création de sociétés de projets locales pour chaque territoire qui déterminera la gouvernance adaptée et nous ne défendons à ce propos que la décision d'intervention de la G P sur les projets proviennent bien d'une demande des collectivités porteuses la région et les M. Ce chantier s'appuiera ensuite sur une expertise partagée entre S N C F Réseau et la S G P avec une répartition des rôles clairs et des discussions avec les exécutifs locaux concernés. La compétence de la G P n'inclura ainsi pas les infrastructures et les installations de service déjà en exploitation afin de tenir compte de son évolution. Le groupe R D P I a souhaité déposer deux amendements et nous en discuterons à l'article Construire Les futurs ermes avec l'ambition exposée précédemment c'est enfin nécessairement entreprendre des investissements significatifs en février dernier la première ministre a également puu annoncer un plan de cent milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici à deux

la déclinaison du plan de financement qui devra accompagner les demandes de labellisation est vous le savez très attendue au delà de la forme du cadre que cela prendra nous partageons la nécessité de solutions partagées à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d'investissement et de fonctionnement,

tiens en conclusion du passer rail qui doit permettre plus d'attractivité afin de rendre possible un choc d'offre accessible qui fait appel à l'intelligence collective territoriale nous voterons ce texte essentiel qui concrétise unembossed qu'il répond à un impératif écologique. Je vous remercie Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Olivier Jacquin, du groupe socialiste, écologiste et républicain pour une durée de 6 min. Mᵐᵉ la Présidente, je suis ravie de reprendre du service sous cette Présidence éclairée M. le Ministre, chers collègues, il y a un peu moins d'un an, alors que nous étions en pleine préparation budgétaire nous apprîmes au détour d'une vidéo que le président de la république décida sur un coup de tate de dployer dix projets de e r métropolitains un nouveau fait du prince un nouvel épisode de l'incohérence complète de la politique qu'il mène en matière de transports depuis deux mille dix sept passant un jour des mobilités du quotidien à la relance de la grande vitesse le lendemain suivie d'un contrat de performance de s n c f réseau qui bloque le ferroviaire et nous voilà revenus à la case départ sans que les étapes précédentes ne soient requiers en serons empêchés aujourd'hui puisque l'article 40 a frappé mon amendement pour réformer ce contrat de performance et mettre fin au carcan de S N C F réseau, alors que le ministre a entamé cet été, des concertations pour bâtir une nécessaire nouvelle loi de programmation des infrastructures et que l'ensemble des acteurs à commencer par les collectivités crient au manque de financement nousmêmes de la création d'une nouvelle offre de mobilité et si je salue le retour de la priorité, mobilité du quotidien à travers ce texte, je pense M. le ministre et sans faire offense au président Zuleeg Zuleeg de loi aurait été plus adapté en plus d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'etat, vous auriez pu plus aisément y accoler un indispensable volet financement et éviter qu'une nouvelle fois nous ne légiférions à l'aveugle puisqu'à l'heure du quarante neuf trois Nous n'avons aucune idée de ce qu'il adviendra de nos avancées lors des débats budgétaires. Mais Simon Husa, mon collègue reviendra sur la question des financements après moi. Je suis, chers collègues, particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cet hémicycle pour parler de mobilité du quotidien dès le début de cette Permettez moi, dès à présent de saluer et remercier le rapporteur Philippe Tabar pour son excellent travail. Il a adopté un esprit tant d'ouverture que de compromis tout au long de ces dernières semaines afin que nous aboutissions à un texte le plus consensuel possible si la moitié d'entre nous était en campagne ces derniers mois toutes et tous nous avons été interpellés sur ce sujet prégnant interpellés sur ce sujet prégnant des mobilités le déploiement des solutions contenues dans la boîte à outils qu'a été la loi d'orientation des mobilités de deux mille dix neuf est en cours encore inachevée nous accueillons donc très positivement cette nouvelle brique dans la boîte à outils elle servira à stimuler les autres en développant de nouveaux services dans une dizaine de métropoles, du moins en l'état actuel du texte et c'est là dessus que je voudrais m'arrêter chers collègues déjà parlementaire ou non, aucun d'entre nous n'a oublié la crise des gilets jaunes et les fractures sociales et territoriales qu'elle a révélées, le danger est grand

déjà mal acceptées et des mesures compensatoires trop faibles et trop lente à déployer. Le groupe socialiste, écologiste et républicain, salue donc le fait que l'assemblée ait décidé, cet été, d'étendre l'intention d'emmanuel Macron en passant de simples projets de réseau express métropolitain à de véritables services express régionaux métropolitains sortant de fait du seul mode ferroviaire. La moitié du chemin est faite allons au bout de la logique si nous voulons être à la hauteur de nos ambitions climatiques nous ne pouvons nous contenter de dix projets dans les plus grandes métropoles osons le choc d'offre comme nous y invite s n c f réseaux depuis deux la note nos grandes entreprises de transport de nombreux présidents de région et d'agglomération ou encore le conseil d'orientation des infrastructures quittons la seule logique métropolitaine pour celle des mobilités pour tous étendons cette belle idée des Cer à des agglomérations de plus petite taille. Elle ne saurait être réservée aux seules métropoles, organisons les déplacements de demain autour d'une offre complète de services en s'appuyant sur les logiques de rabattement depuis la voiture individuelle socialisée par le covoiturage, l'autopartage et le vélo v.. Les transports plus lourds. Le bus à haut niveau de service et les trains accompagnons les collectivités périurbaines pour offrir des solutions aux habitants qui seront demain exclus des et pour qu'ils puissent continuer de venir travailler étudier et accéder aux services publics quii ont souvent disparu de leur environnement immédiat à commencer par les professionnels de santé bien sûr et nous y reviendrons longuement. Le ferroviaire doit avoir une place prépondérante dans cette organisation et rester quand il existe l'épine dorsale de l'écosystème de mobilité. Nous aurons les débats concernant la transformation de la société du Grand Paris. et les garanties apportées à S N, C F, réseaux comme à Gare et Connexions, ainsi qu'à leurs salariés, nous aurons les débats techniques concernant les pactes de gouvernance avec les collectivités, la planification et la labellisation l'interopérabilité ou encore les contrats opérationnels de mobilité mais je veux profiter de cette discussion générale pour vous enjoindre à travers cette proposition de loi bienvenue mais encore incomplète a posé les bases d'une grande politique publique de mobilité qui n'oublient aucun territoire et encore moins, la nécessaire transformation de nos déplacements face à l'urgence climatique, faisons confiance à nos régions et à intercommunalités.

avait massivement contribué. Alors Alors, allons y, je vous remercie Cher collègue. La parole est maintenant à M. Didier Mandela, du groupe Les Républicains, pour 7 min. madame la présidente monsieur le ministre monsieur le président de la commission monsieur le rapporteur cher philippe mes chers collègues je me que la présente proposition loi traduise enfin les ambitions affichées dans la loi d'orientation sur la mobilité promulguée fin deux mille dix neuf de saturer les villes et leurs accès améliorer les liaisons entre les liaisons entre les territoires ruraux périurbains et les pôles urbains telles étaient les priorités de la loi d'orientation des mobilités portée par la ministre d'alors elisabeth borne je vous souhaite la même trajectoire, M. le ministre et dont j'étais rapporteur pour le Sénat. Pour mémoire, la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'état fixée par cette loi qui visait notamment à réduire les inégalités territoriales, renforcer l'accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, ainsi que les offres de déplacements du quotidien. L'un des cinq programmes d'investissement portait sur la résorption de la saturation des grands œufs ferroviaires, avec pour objectif le doublement de la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains. Malheureusement, ainsi que nous l'avons exposé à maintes reprises dans cet hémicycle, l'exécution de cette loi a confirmé les craintes que nous avions exprimées en commission mixte paritaire de manière générale les investissements, n'ont malheureusement pas suivi et la régénération du réseau ferroviaire n'av pas encore eu lieu après quatre ans et plusieurs annonces du président de la République n'ont suivi d'effets Nous devons ce texte à une initiative parlementaire du Président, en l'occurrence de la commission de l'énigme loppement durable de l'assemblée nationale, jean marc zulia amicalement la mise en place des services express régionaux métropolitains est réclamé par les élus locaux depuis de nombreuses années dans la plupart des métropoles les projets existent mais peinent à se mettre en place mille dix neuf jean baptiste djem affirmait dans ce même dans ce même hémicycle en matière ferroviaire il s'agit de doter les métropoles de liaisons transversales rapides fréquentes et interconnectées à l'image du réseau express régional de france La présente proposition de loi va plus loin car si les Serbes s'appuient sur le renforcement des dessertes ferroviaires, il s'agit, avant tout, d'offrir aux usagers une offre multimodale de transport collectif public. une offre multimodale qui va intégrer plusieurs modes de transport tels que le covoiturage, l'autopartage ou encore les réseaux cyclables, à l'initiative de la Commission et de notre rapporteur plutôt que d'interdire contraindre et sanctionner donnons aux usagers les moyens de préférer un mode de transport réduire les inégalités et inscrire les territoires et leurs usagers dans la transition écologique, c'est tout l'enjeu des nouvelles mobilités la présente proposition de loi doit permettre de donner corps et de soutenir ces initiatives locales. C'est bien de cela, dont il s'agit accompagné des projets adaptés aux territoires à cet égard. je remercie l'excellent rapporteur, Philippe Tabou. Par, ailleurs, il est important de le souligner membre du conseil d'administration de la I T et du conseil Conseil d'orientation des infrastructures. Les Serbes doivent être, je le cite,

aussi à l'initiative de notre rapporteure. Nous avons avec mes collègues membres de la commission d'aménagement du territoire et du développement durable notamment souhaité inclure une consultation systématique des maires et des départements en amont. et renforcer les procédures et renforcer le rôle de la région Nous espérons que le gouvernement soutiendra ces modifications qui participeront, j'en suis certain, au succès des projets, Le texte transforme la société du de Grand Paris en société des grands projets et lui en confie la maîtrise d'ouvrage. Il est rassurant que l'ensemble du territoire puisse bénéficier de l'expertise de cette société qui a qui conduit le chantier du Grand Paris Express chantier pharaonique, cela a été évoqué, qui, rappelons le, a été primé par l'université de Harvard, en début d'année. Pour autant, les projets qui seront déclinés dans les territoires ne vont pas bénéficier des mêmes facilités infrastructures que le Grand Paris Express. Express président nous l'a confirmé il n'y a pas de réplicabilité du modèle économique. Soyons lucides si les projets initiés par les élus locaux n'aboutissent pas, c'est bien souvent en raison d'un manque de financement. Plusieurs pistes ont bien été évoquées emprunt, fiscalité, Pété appropriation foncière tout cela pouvant être mixé évidemment, mais la question n'est pas tranchée, ce qui est certain, c'est que l'état doit prendre sa part. Sauf à aggraver les inégalités territoriales les serbes ne peuvent pas concentrer l'ensemble des finances locales dédiées aux transports et à la mobilité à l'instar de ce qui s'est produit avec le g

à comparer aux deux six milliards prévus dans la loi d'orientation des mobilités avec une prise en charge de l'état c'est ce qui était intégré à hauteur d'un virgule trois milliards cette somme semble très éloignée des treize milliards d'euros chiffrés en juillet deux

Ainsi modifié, et avec des réserves évidemment, sur le volet du financement, le groupe Les Républicains soutiendra cette proposition de loi. Chers collègues. est donc maintenant à M. Simon Husa, du groupe socialiste, écologiste et républicain pour 3 min

pour autant comme l'a rappelé Olivier Jacquin, nous ne saurions nous en contenter et c'est pourquoi nous proposerons de rebaptiser les ser ms en service express régionaux de mobilité en effet qu'il s'agisse de l'enjeu écologique avec l'objectif dans le secteur des transports de vingt huit de décarbonation à l'horizon deux mille trente par rapport à deux mille quinze ou encore des enjeux territoriaux et sociaux dans le contexte d'inflation forte et de renchérissement très net des prix de l'énergie la massification des transports collectifs y compris sur la partie ferroviaire constitue désormais un impératif politique qu qui nee doit oublier aucun territoire. Nous le savons bien et les travaux de notre commission l'ont rappelé avec insistance, le nerf de cette bataille capitale pour rendre toujours plus accessibles les mobilités décarbonée est avant tout financier or sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres il y a malheureusement monsieur le ministre loin de la coupe des promesses aux lèvres de la réalité entre l'annonce des cent milliards d'euros d'ici deux mille quarante pour la nouvelle donne ferroviaire et les huit cents millions d'euros pour les serbes sans oublier les besoins de régénération d'un réseau ferroviaire particulièrement dégradé le fossé est béant sur les fermes cela a déjà été dit nous sommes sur les cinq prochaines années à peine dix pour cent de l'effort en intégrant les financements des régions le rapport de l'autorité de régulation des transports de juillet deux mille vingt trois est par ailleurs particulièrement inquiétante sur l'avenir de notre réseau ferroviaire le président par intérim notre ancien collègue philippe richer écrit ainsi

des dépenses de régénération qui décroissent depuis deux mille seize inférieure de vingt cinq en préconisations une concentration des moyens sur le réseau structurant le pluss circulé tout cela préfigure une néfaste archipélagique aggravation des disparités territoriales pour cela nous serons donc vigilants à ce que le déploiement des termes n'absorbe pas tous les financements et ne se fasse pas au détriment de l'indispensable modernisation du réseau. Si nous voulons être collectivement à la hauteur des défis de la régénération et du développement des mobilités décarbonées pour lesquelles le ferroviaire et l'épine dorsale, nous devons en effet d'urgence revoir un système de financement des mobilités à bout de soufflet

des les recettes fiscales dédiées et sur le M a la suppression du plafonnement, un M a différencié en fonction des projets et des bassins de mobilité afin de permettre des développements d'offres de transports multimodales ciblés par territoire.

quoi qu'il en soit. le texte de la Commission comprend de nombreuses avancées qui vont dans le bon sens. Nous voterons donc ce texte, je vous merci beaucoup, chers collègues, la générale est close, M.. le Ministre, quelques mots avant de passer à la discussion du texte de la commission

d'abord même si ce n'est pas l'objet de cette proposition de loi de débat de la question des financements j'entends un certain nombre d'interrogations sur l'investissement global dans le ferroviaire je ne le paierai pas intégralement nous aurons l'occasion de parler

Les crédits annuels consacrés aux mobilités dans dans les mandats que nous sommes en train de déployer et de négocier avec chacune des régions avec un effort qui est cohérent et ciblé parfois c'est d'ailleurs critiqué parce que c'est un choix courageux nous réduisons en effet la part consacrée réduisons en mais pour augmenter massivement y compris pour faire place à ces fameux huit cents millions d'euros la part consacrée au ferroviaire et aux transports publics à prendre deux tiers de chacun des mandats adressés par la première ministre à nos préfets de région pour discuter avec les premières régions c'est un effort conséquent le réseau ferroviaire nous aurons l'occasion d'en discuter et de le matérialiser nous avons fait un effort important l'an dernier nous allons faire une marche massive supplémentaire dès l'an prochain et c'est un engagement qui sera je vous rassure gravé dans le marbre de la première ministre présenté sur le fondement du rapport du e i d'augmenter de cinquante d'ici deux mille vingt sept les crédits annuels consacrés à notre réseau ferroviaire car oui en effet vous l'avez dit sur les différents bancs dans les différentes interventions le point de faiblesse français en matière de ferroviaire c'est le réseau et l'âge du réseau ont réinvestit je regrette que cela n'ait pas été fait plus tôt mais nous réinvestissements massivement je nee cherche pas la polémique mais ce sont des chiffres vérifiables ensuite sur les fameux sept cent millions d'euros devenus huit vous montre le chiffre exact il est de sept cent soixante sept millions d'euros et c'est le chiffre qui est en entrée de discussion je ne devrais pas dire ça en bon budgétaire en entrée de discussions avec chacune des régions et mesdames et messieurs les sénateurs j'entends votre interpellation mais je me permets de la répercuter aussi certains la connaissent personnellement aux représentants des régions cent soixante sept millions d'euros vous me permettrez de les arrondir à huit cents qui augmenteront peut être un petit peu en cours de de négociation soit avec en face des crédits similaires de la part des régions je pense que ce sera le cas j'espère que ce sera le cas mais si on additionne les deux et donc c'est un effort conjoint vous m'aurez compris que nous devons porter ce sera ce sera déjà plus d'un milliard cinq cents millions d'euros pour une première étape j'insiste et c'est ensuite sur le fondement de la loi qu'on discute ce soir que les plans de financement serme par serme seront présentés et à ce moment là vous pourrez d'ailleurs le vérifier en toute transparence il faudra évidemment que l'état soit au rendez vous comme il faudra que les collectivités soient au rendez vous et comme pour ceux qui le souhaitent pour les collectivités qui le souhaitent des ressources fiscales dédiées ce n'est pas une obligation c'est une faculté pourront être mobilisées c'est là que nous verrons évidemment le coût et le plan de financement et d'investissement de chacun de ces services express régions métropolitains mais admettez que pour une politique qui se met en place et qui commence huit cents millions d'euros en train de négociation c'est un ticket d'entrée qui est pas totalement indécent il va augmenter il va être euh matcher si je peux le dire en mauvais français par les régions je l'espère bien et il va être ensuite affiné en cours de déploiement de ce service express régionaux métropolitains je rappelle qu'en parle en plus de la première étape vingt sept et pour beaucoup de projets ce sera une phase d'études je l'espère de travaux aussi mais d'abord d'études donc on ne parle pas de sommes qui sont ridicules j'insiste loin de là avec un engagement très clair de l'état donc j'attends qu'il soit

donc nous irons ensuite qui est indicatif je l'ai dit pas au sens où je néglige ces montants mais au sens où par définition puisque ces montants viennent des territoires vers l'état et ces projets sont portés par les collectivités soumis à l'approbation de l'état c'est ensuite à partir du premier semestre de deux mille vingt quatre sans doute que l'on définira et détaillera les plans de financement l'état sera au rendez vous mais évidemment il faut que les collectivités soient aussi au rendez vous et il faut aussi ce sera encore une fois volontaire et au cas par cas que l'on ne s'interdisent pas les ressources fiscales dédiées et affectées on l'a fait pour la série du Grand Paris. cela peut être une solution pas forcé mais possible pour différents projets de service express, région métropolitain Je voulais apporter le Ministre, nous

Mᵐᵉ la Présidente, M. le ministre, MM. le rapporteur et le Président de la Commission, mes chers collègues, Si les Français sont prêts à réduire leur recours à la voiture. Encore faut il que nous leur proposions des alternatives pratiques et acceptables. La présente proposition de loi y répond en prévoyant la création de services express régionaux métropolitains. ci ont en effet la double ambition de proposer des services de transport collectif qui faciliteront la vie de nos concitoyens tout en permettant d'accentuer la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un secteur des transports, qui en aimait encore beaucoup. Je tiens également à saluer le travail de fond sur ce texte de notre collègue rapporteur, Philippe Tabar, de celui celui de mes collègues de la commission du développement durable. ont permis de l'enrichir de manière significative, rien que sur l'article 1ᵉʳ. Leurs amendements ont permis d'insister sur l'importance de promouvoir une offre de mobilité multimodale. Ils ont aussi rappelé rappelé la nécessité de penser les Serbes à partir des territoires en incluant autant que possible les collectivités en amont de leur déploiement. Je me réjouis enfin que le gouvernement mette un coup d'accélérateur sur ses services dans le siège des annonces récentes du président de la République. Je compte sur vous, M. le ministre, pour que l'état soit au rendez vous. Ces projets sont attendus avec impatience dans beaucoup de métropoles mais aussi bien au delà dans les Pyrénées Atlantiques, par exemple le projet de E R pyrénéen apporterait beaucoup car les dessertes ferroviaires sont aujourd'hui de piètre qualité avec à la fois peu de chers collègues nous

madame la présidente pour ce tout premier amendement nous proposons de renommer ce texte en lui enlevant le qualificatif de métropolitain pour le remplacer par services express régionaux de mobilité. Il faut le comprendre comme un point d'enthousiasme de notre part par rapport aux logiques de mobilité du quotidien. Le texte a été bien amélioré par la Commission en conjuguant intermodalité et multimodalité sur base ferroviaire et routière essentiellement Et Il nous semble que cette proposition permettrait d'améliorer son acceptation car si le S E R métropolitain pourrait encore accentuer la fracture territoriale, le S E R mobilité vise au contraire à généraliser le concept de densification et à rendre ces services de mobilité accessibles à toutes les strates de l'urbain là où la demande de transport est est importante, etc, en sortant d'un métropolitain trop restrictif quatre ans après la crise des gilets jaunes et alors que se mettent en place les zones à faibles émissions mobilité dans les principaux pôles urbains du pays, qui vont compliquer l'accès des habitants en périphérie il est plus que jamais temps d'accélérer le déploiement de toutes les solutions de mobilité alternative à la voiture individuelle émettrice de gaz à effet de serre et particules fines sans renforcer toujours l'avantage le e métropolitain déjà

Il faut que la multimodalité soit efficace et fluide, il est donc essentiel de privilégier un usage facilité, clair et simple pour les simple pour les usagers des services de billet, étique et d'information. Donc, il faut prendre en compte les attentes des usagers qui ont besoin de mobilité quotidienne. fluide, pratique je le disais tout à l'heure et quii se fiche des prés carrés de nos différentes collectivités et donc le texte en commission la Commission proposait de supprimer abruptement la nécessité d'aller v. une biotique intégrée. Ce que nous proposons, c'est de le réintégrer de façon pragmatique il ne s'agit pas de charger la barque des projets Serm le mieux et parfois l'ennemi du bien. Et donc, il s'agit c'est la formulation de cet amendement non plus de garantir mais de permettre donc on ne soit pas obligés d'assurer l'interopérabilité pour avoir droit au label Ser Mes et aux financements qui vont bien avec, mais on mettra en place des conditions qui le permettront. Merci, quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur sur ces deux amendements pense qu'il y a y a un petit problème concernant jacques fernie sur sur cet amendement je pense qu'il a défendu plutôt l'amendement seize rectifié au lieu du dix sept rectifié

en coopération avec la région, de consulter systématiquement chaque maire des territoires impactés. Cette disposition pas franchement inspirée par la confiance sur la faculté de l'intercommunalité centre de la métropole à conduire à piloter à sa façon spécifique la démarche partagée de ce projet de territoire donc faisons leur confiance et nee réduisons pas ses projets à la somme de préoccupations strictement communales

l'inscription des métropoles dans l'expression erb les encouragent à s'impliquer dans ces projets En outre, loin d'opposer les métropoles aux autres territoires le nom de E M leur confère au contraire une responsabilité sur les mobilités au delà de leurs limites strictes. Enfin, je ne pense pas qu'il soit réaliste pour le moment de décliner le modèle de des sermur tout le territoire l'urgence c'est pour l'instant de le déployer autour des métropoles mais c'est un débat qu'on va avoir dans quelques instants concernant donc je vous propose un avis défavorable sur cet amendement vingt huit quant à l'amendement dix sept je partage l'intention louable de ces signataires d'alléger la procédure de lancement des serbes toutefois je maintiens comme je l'ai dit la semaine dernière que consulter les maires en amont du déploiement des serres me semble d véritablement essentiels je donnerai un avis défavorable à l'amendement merci

pas concurrents mais complémentaires, qu'il faut encourager aussi à travers ce texte et ce seront les principales collectivités porteuses de ces projets sur leur territoire. Donc, je pense qu'il est important qu'on garde cet équilibre entre ces deux niveaux de collectivité j'en profite pour souligner parce que c'est un point euh non pas technique mais politique essentiel quand on parle de E r métropolitain comme on l'a fait au départ ou de services expressément métropolitains, ça n'est pas métropolitain ça n'est pas métropolitain au sens du cœur de ville. J'insiste beaucoup là dessus et toutes les collectivités qu'ont commencé à déployer ou à travailler sur ces projets je crois peuvent en témoigner le partage pour répondre d'ailleurs à la première intervention c'est justement pour apporter des solutions alternatives à la voiture monsieur le sénateur pour des gens qui voudraient avoir des solutions alternatives mais qui n'en ont pas qui sont à trente cinquante ou quatre vingts kilomètres des centres villes c'est pour ces personnes là ces français là cess automobilistes parfois contraints que nous proposons d'avoir

d'alternative à la voiture individuelle aujourd'hui et qui voudrait à la fois pour des raisons écologiques et de pouvoir d'achat en même temps voilà donc je préfère qu'on garde le mot métropolitain par l'autre train un tout petit peu long je serais plus court après sur ce premier amendement sur le dix sept rectifié je suis si je puis dire agnostique je partage l'idée il est forcément particulièrement sensible et attentif qu'il y a évidemment une consultation des maires c'est indispensable mais je crois que ça naturellement dans la pratique je ne suis pas sûr qu'il faille formaliser cette étape

qui vote contre qui s'abstient et n'est pas adopté l'amendement dix sept un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement qui vote pour

Mᵐᵉ la Présidente, M. le ministre. Chers collègues, donc cet amendement vise, dans la continuité de mon intervention en discussion générale, à mettre l'accent sur la prise en compte de l'état général de notre réseau On a pu dire On a pu dire les uns les autres au cours de cette discussion générale, à quel point, euh, ce réseau était particulièrement vieillissant quand on compare aux autres pays européens proche de nous. La comparaison est d'ailleurs assez terrible, que ce soit en termes de régénération ou d'équipement au regard des obligations qui nous sont faites. sur le plan européen, et ce vieillissement du réseau a un impact évidemment direct sur la qualité du service rendu à nos concitoyennes et nos concitoyens. L'enjeu, pour nous, ce n'est évidemment pas d'opposer les uns aux autres les serme à la régénération mais faire en sorte que cette dernière soit bien prise en compte hors le contrat de performance dont nous avons parlé qui est fondé sur la règle d'or limite de fait la capacité d'investissement de s n c f réseau et l'on voit bien que les chiffres ne sont pas au rendez vous monsieur le ministre parce que seize et c'est l'autorité de régulation des des transports qu'il écrit ce n'est pas nous les dépenses de régénération sont en baisse constante et donc il y a là un signal d'alerte et d'ailleurs le scénario tendanciel retenu par l'a r rt confirme bien là aussi cette dégradation annoncée

dix fois cette même enveloppe et l'on voit bien le risque à venir celui d'une archipelago où on aurait des parties du réseau ferroviaire très bon état et d'autres extrêmement dégradés nous souhaitons garantir l'équité et la qualité de service pour l'ensemble de nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est l'objet de cet amendement. Je vous remercie, Oui, chers collègues, le le Le but légitime de votre amendement, c'est de veiller à ce que on ait une bonne connaissance de l'état du réseau et notamment du problème du vieillissement. C'est quelque chose qu'on partage et je peux que souscrire aux propos que vous avez tenus sur sur ce réseau, pourtant cet amendement me semble pleinement satisfait par les études préparatoires et la mise en place des termes qui vont permettre, dans les faits, de réaliser ce diagnostic d'autre part, surtout le texte de la Commission prévoit, grâce à l'ajout en commission justement d'annexer aux contrats de performance à n c f réseau son programme annuel d'investissement qui permettra d'établir ce diagnostic,

Merci M. le ministre, sur cet amendement. même avis, euh, avec les mêmes arguments, Mᵐᵉ la Présidente, s'il s'agit de faire un diagnostic, je crois que cela est traité par le diagnostics préalables systématiques et les études qui seront réalisés avant le déploiement des Ser Mes comme l'indiqué M. le rapporteur s'il s'agit d'avoir une préoccupation plus générale pour l'état du réseau, l'investissement ou le réinvestissement nécessaire dans le réseau, je le partage absolument, je crois que ce n'est pas dans le cadre des R R Mes qu'il faut le traiter spécifiquement, c'est dans le cadre du débat budgétaire que nous aurons, c'est dans le cadre du contrat de performance que nous actualiserons, mais je partage la préoccupation simplement je suis aussi vigilants à ce qu'on n'alourdisse pas les procédures, il y aura des études et un diagnostic préalable, de toute façon et le débat général sur l'état du réseau, je crois que nous l'aurons dans un autre cadre.

très clairement pour remettre sujet, euh sur le dessus de la pile. Donc on regarde des éléments apportés par M. le rapporteur et par M. le ministre, nous retirons cet amendement. ci. beaucoup, chers collègues, nous poursuivons par l'amendement 50 présenté par M. Jacquin,

taille de strate urbaine par celui de cinquante pour permettrez à des étoiles ferroviaires de plus petite dimension de développer le système des Ser Ms dans le même souci de généralisation que j'ai

Oui, Mᵐᵉ la présidente, chers collègues, euh. soyons réalistes, il n'est pas possible de, pour le moment, de décliner le modèle des Serbes sur tout le territoire. Il est particulièrement ambitieux. Cela ne signifie pas que les espaces ruraux périurbains n'ont pas vocation à bénéficier des transports collectifs de qualité Et puis vous savez que je suis un ardent et un farouche partisan des petites lignes ferroviaires. Je l'ai dit plusieurs fois, et j'ai proposé un certain nombre d'amendements sur ce sujet dans ce même hémicycle dans ce même hémicycle, mais je crois que le texte que nous avons abordé aujourd'hui euh doit rester sur un sujet bien particulier, qui est celui des services express régionaux métropolitains et donc je pense que cet amendement ne ne colle pas à ce qui est prévu dans ce texte, je vous demande de le retirer ou sinon j'émettrai un avis défavorable tout en entendant les arguments dont vous faites part sur la mobilité sur l'ensemble des territoires. M. le rapporteur, Avis du Gouvernement. oui le même avison les termes sont essentiels et ne sont pas exclusifs de tous les outils de mobilité je pense notamment à ce que nous déployons à travers les annonces qu'a faites mme ma collègue chargée des collectivités locales où nous déploierons quatre vingt dix millions d'euros sur les solutions de mobilité rurale pour les territoires plus petits en complément d'autres outils

pour une série d'agglomérations, toutes celles que j'ai rencontrées, qui m'ont sollicitées d'une façon ou d'une autre, à court ou à moyen terme pour leur projet, sont aujourd'hui éligibles avec les critères actuels, donc je crois que nous avons ici un bon équilibre, donc défavorables à cet amendement. Merci beaucoup. Je oui, je vous en prie, M. Jacquet. J'ai bien entendu M. le rapporteur, M. le Ministre, votre explication on ne vise pas à régler toutes les questions du ferroviaire par cet amendement, on vise à le rendre possible le serme pour des collectivités de plus petite taille et on n'est pas dans le rural il s'agit pas des petites lignes ferroviaires c'est une ville de trente mille habitants qui a une étoile ferroviaire peut lancer le même modèle de serbe si elle en a la volonté politique c'était ça l'ambition et la précision que je voulais apporter l'amendement est bien évidemment maintenu chers collègues je vais donc mettre aux voix cet amendement avec deux avis défavorables de la commission et du gouvernement Gouvernement qui votent contre. qui s'abstient n'est pas adopté Continuons la discussion avec quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune, M.. Barros, pour l'amendement numéro quatre. Mᵐᵉ la Présidente, M. le Ministre, chers j'ai fernie tout à l'heure, ouvert un peu la voie. Donc on va on va poursuivre la discussion ensemble dans la version qui nous est parvenue initialement. Le texte prévoyait une interopérabilité des services d'information des voyageurs et également des billets

on peut par exemple souligner les difficultés rencontrées par de France mobilité en Île de France avec la fin du ticket papier remplacé par une carte réutilisable qui ne fonctionne pas sur les réseaux Ee R. Il faut donc un ticket papier pour le E R et une carte magnétique pour le réseau lorsqu'on n'est pas abonné Cela risque d'être aussi la même chose pour le grand Paris Express. Notre objectif avec cet amendement est d'éviter aux usagers d'avoir le sentiment de passer d'un réseau à un autre lors d'un même voyage et de passer trop de temps au distributeur de titres de transport. Je vous invite à faire l'expérience Ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus a de plus efficace dans la vie. C'est la même chose en matière d'information des voyageurs où il y a besoin d'avoir une information mutualisée surtout sur un réseau où différents opérateurs peuvent être présents. présent. Nous souhaitons que cette mesure d'interopérabilité s'applique par la création d'un billet unique. Nous ne sommes pas allés jusqu'à proposer un tarif unique désolé mais c'est aussi V. cela qu'il faudra attendre pour favoriser l'utilisation des transports en commun pour, en tout cas, on veut que cela fonctionne. Chers collègues, bien, nous continuons avec trois amendements identiques. On commence par le numéro huit avec M.. Rochette.

facilitant effectivement l'avis des voyageurs et de tous les utilisateurs de de de ces réseaux futurs Serm en en réintroduisant les notions effectivement d'interopérabilité et d'interconnexion à la fois à la fois des systèmes d'information voyageurs mais également des systèmes billettiques, tout en remplaçant également le rôle de la région en tant qu'autorité organisatrice de mobilité et globalement, en respectant les équilibres de chacune

ça vous va très bien. alors je vais donc mettre ces quatre amendements en demandant l'avis de la Commission sur le numéro quatre et ensuite sur les trois identi. je vous en prie, M. le rapporteur. L'amendement quatre semble, pour l'heure, source de complexité. les O M travaillent depuis de longues années à assurer une meilleure interopérabilité de la bie bie éthique ce sont des années de travail sur des sujets très complexes aux enjeux tant techniques que politiques et financiers ne donnons pas un coup de pied dans la fourmilière en imposant la création immédiate d'un billet unique pour les différents modes de transport collectif inclus dans les Serbes Serbes, Cela pourrait ralentir malheureusement leurs lancements. Cela Tant j'entends parfaitement votre souhait que le texte fasse référence à cette question de l'interopérabilité et de la billettique. c'est pourquoi la Commission sera elle favorable aux amendements huit rectifiés, 11 rectifiés, 16 rectifiés,

corrobore les avis du rapporteur

on va pas ouvrir le débat ici. Mais le phénomène de métropolisation, Euh l'accaparement euh euh de plus en plus d'emplois. Et et le l'éloignement euh, de, de l'emploi et du domicile font que, effectivement, on a de plus en plus de de nos concitoyens qui sont amenés à changer finalement de secteur et à donc à être confronté à toute cette problématique. Il nous semble cependant et pour en avoir discuté que, bien évidemment, l'objectif, c'est que ça avance que tout ceci puisse se donc nous nous acceptons la proposition faite par M. le rapporteur, nous allons retirer notre amendement, bien évidemment soutenir les suivants, mais mais vraiment j'insiste pour que l'on puisse et avancer pas pour avoir une carte qui marque l'identité régionale mais pour avoir effectivement une capacité en matière de billettique qui facilite euh les déplacements, la visibilité, y compris financière, de ce que cela, Euhh implique Euh et et je n'en doute pas, en tout cas, pour les usagers une une meilleure rentabilité de leurs déplacements. Mᵐᵉ la Présidente, Coker Man, donc je considère que l'amendement quatre est retiré. Je vais donc pardon M. Jacquin

nous avons écrit un peu plus légère, plus souple parce que, en commission, on avait été sensibles aux arguments du rapporteur mettant en avant le chef de fila régional et considérablement les procédures nous voterons pour les les amendements qui ont reçu un avis favorable et qui feront tomber le note, mais on arrivera au même résultat je vous remercie cher collègue plus d'explication de vote je vais donc mettre aux voix monsieur le rapporteur pardon je vous en prie Oui, excusez moi, j'ai une bonne nouvelle pour le sénateur Jacquin son amendement ne tombera pas, donc il pourra le défendre, il aura un avis favorable, il est complémentaire, voilà je vais mettre aux voix chers collègues trois amendements identiques qui ont fait l'objet de deux avis favorables qui votent pour qui vote contre, qui s'abstient, ils sont donc adoptés. Nous continuons avec l'amendement 12 c'est Mᵐᵉ Guillotin qui défend. Je vous en prie.

donc c'est un amendement de M. Cabanel que je présente c'est en fait le but, c'est qu'aucun territoire ou aucune commune ne soit soumise à une aire d'un pôle majeur d'emploi et de population autour duquel se structure interne ne doit être oubliée, que ce soit dans un processus de concertation initiale ou dans un déploiement. Affectif Tif Les travaux en commission ont permis effectivement de responsabiliser et de concerner davantage les collectivités territoriales, notamment les communes affin, qu'un projet d'une telle ampleur et d'une telle dimension ne puisse faire sans l'avis des maires il ne serait pas souhaitable non plus que certains d'entre eux en soient délaissés afin que le maillage territorial des futurs termes soit réalisé sur des critères sur des critères objectifs cet amendement propose donc de baser le périmètre du e m sur le zonage en aire d'attraction des villes développé depuis deux mille vingt par l'insee en fait le zonage en aire d'attraction des villes est une approche zonage en aire d'attraction est également une maille d'étude adaptée à l'analyse des réseaux de travailleurs pendulaires entre d'économies, d'entreprises et d'individus en interaction. Voilà en fait Il nous semble important donc, si le développement d'un service Euh express régional métropolitain a pour but le désenclavement des territoires périurbains et ruraux par un choc d'offres multimodales autour des métropoles et grandes agglomérations, il semble important d'établir ce périmètre rigoureux et objectif permettant également d'éviter une aspiration des financements parés pour les métropoles, auquel cas la principale cible du texte pourrait être manquée. chers collègues, est l'avis de la commission sur cet amendement. Mᵐᵉ la sénatrice, malgré les la conviction que vous avez mis à défendre cet amendement, je vais vous donner quand même un avis défavorable, si vous nee le retirez pas. mètre du déploiement des Serm proposé dans cet amendement est pertinent lorsqu'on réfléchit de façon générale au périmètre d'un cependant faire de ce périmètre qui pourra opportunément servir de base indicative un périmètre prescriptif me semble excessif parfois compte tenu des dynamiques locales, l'inserm pourra aller par exemple au delà de l'ère d'attraction de métropole. le cadre proposé par cet amendement est trop rigide. fusc confiance aux acteurs locaux pour élaborer le périmètre le mieux adapté à leur situation. Avis défavorable ou je vous propose un retrait préalable peut être Merci, M. le rapporteur, Avis du Gouvernement sur cet amendement. Mᵐᵉ la sénatrice, ne m'en voulez pas à travers vous le sénateur Cabane, mais je serai obligé d'exprimer la même position nuancée mais néanmoins position nuancée mais néanmoins pas totalement enthousiaste de que celle du rapporteur, en vous demandant le retrait et à défaut en exprimant une position défavorable

précieuse les uns les autres au cours de nos différentes interventions. Les mobilités sont devenues un sujet de préoccupation majeur, quotidien pour nos concitoyennes et nos concitoyens, c'est important de pouvoir leur donner la parole dans le cadre de ces projets structurants et c'est l'objet de cet amendement, prenant appui sur des initiatives qui ont déjà été mis en œuvre dans un certain dans un certain nombre de régions. encore une fois nous ne découvrons pas la concertation les uns les autres. Il est évidemment essentiel d'associer les élus, mais de nee pas oublier nos concitoyennes et nos concitoyens. merci chers collègues, habit de la Commission. C'était un avis favorable pour le sénateur Jacquin, mais on va le conserver également pour vous, chers collègues. Pour les raisons qui ont été évoqués, vous avez rappelé les associations d'usagers

Je pense qu'il est bien de le faire également dans ce cadre là. donc c'est la raison pour laquelle je donnerai un avis favorable M. le rapporteur du gouvernement. Mᵐᵉ la Présidente, je suis sensible à cet amendement Par souci de cohérence, je dirais que je pense que beaucoup de ces étapes seront naturellement prévues par les élus dans la définition des services express régions métropolitains. Il ne faut Il ne faut pas trop formaliser les choses. Néanmoins, il n'est jamais une mauvaise idée de consulter les associations d'usagers, d'entendre pardon leurs avis et leurs remarques puisque c'est pour eux que tout cela est fait. Donc je m'en est fait. Donc je m'en remettrai à la sagesse. bien. Bah écoutez un avis favorable de la commission est un avis de sagesse du Gouvernement, qui vote pour

dans la situation particulière où deux métropoles seraient à proximité. Nous aurons prévu de de fixer cette proximité à 100 km l'une de l'autre la mobilité étant une science globale et connectée, nous demandons par le biais de cet amendement aux collectivités. en proximité de travailler ensemble, et non pas dos à dos, ce qui nous semble être, finalement, une une une proposition plutôt logique et euhh, pleine de bon sens. Mais maintenant, je laisse l'hémicycle en décider. Cher collègue, avis de la commission sur cet amendement. On est toujours sensibles au bon sens. dans cet hémicycle, chère collègue, Mᵐᵉ la Présidente D. Donc c'est la raison pour laquelle on donnera un avis favorable en précisant bien que Et les termes de votre amendement sont importants. qu'on prévoit la faisabilité et l'opportunité de concevoir et de réaliser leurs serm ensemble pour une approche territoriale globale. Voilà, j'imagine que vous avez une petite idée derrière la tête concernant peut être deux, deux métropoles,

c'est deux métropoles à moins de 100 km qui sont Lyon et Saint Étienne et c'est un cas d'autant plus particulier en matière de transport hors ile de France, c'est que c'est la ligne aujourd'hui y compris euh e r euh qui existe et qui est la plus utilisée euh hors de l'île de France une ligne une ligne euh, sur laquelle je reviens pas une ligne, bien évidemment historique, avec des contraintes euh, y compris géographiques, de la proximité d'une rivière, d'un encaissement en fond de vallée du Gier. de nombreux retards, y compris le plus souvent impactés par par l'obligation de desserte et de régularité g v passant par la gare de lyon pardieu et tout ceci transportant pour autant des milliers de de de personnes quie comme la plupart des usagers d'ailleurs

mais pour autant, la réalité et le pragmatisme nous invitent là tout de même, non pas à contraindre mais à bien s'assurer que, effectivement, il y ait travail conjoint, il y est volonté commune et pas simplement d'attendre que chacun s'entende pour trouver une réponse mais parce que nous avons un défi et nous avons un défi, y compris en matière d'aménagement du territoire. c'est C'est que, comme je le disais initialement, c'est la ligne hors île de France qui est la pluss fréquentée quotidiennement.

effect. Cette situation très particulière concerne bien entendu la métropole lyonnaise et la métropole stéphanoise, c'est un amendement qui nous tient très à cœur mais qui peut s'appliquer aussi à d'autres secteurs géographiques que Ronal Ppes, uniquement merci. merci. cher collègue monsieur devina pour explication oui merci madame kicker man je vais rend partager ses son point de vue mais cela dit je trouve cet amendement pour rhône alpes auvergne extrêmement intéressant

Alpes Cher collègue, il n'y a plus d'explication de vote bien je vais donc mettre aux voix cett amendement, qui a eu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il est adopté l'amendement quarante huit présenté par m jacquin la présidente en en commission nous avons fait progresser le en intégrant directement les notions de covoiturage et d'autopartage je vous propose d'aller plus loin en séance en évoquant dans le texte la création de lignes de covoiturage Express, c'est en fait du covoiturage plus très très organisé qui consiste à renforcer les flux sur certaines routes d'augmenter leur fréquentation et de donner plus de chance au covoiturage C'est une technique de covoiturage qui est expérimentée un peu partout en France ces dernières années, notamment par la startup Cov, et qui peut donner de très bons résultats dans le périurbain et avec des coûts extrêmement faibles il s'agit de mieux remplir les les les les voitures existantes et de lutter contre l'auto solistes intégrer cela dans le texte donnerait une chance nouvelle au covoiturage. je tiens à dire que, sur certains territoires, c'est la technique la plus mise en œuvre comme palliatif à l'auto soliste et lorsqu'on n'a pas la capacité à remplir des bus, des niveaux de bus, de cars, express. Ces techniques de ligne de covoiturage express sont une excellente alternative pour les territoires périurbains je vous remercie.

qui prévoit d'ores et déjà l'obligation en cas de déplacement d'un serme d'examiner la faisabilité et l'opportunité de convertir une section d'autoroutes ou de voie express à trois voies en une voie réservée au covoiturage au transport collectif, mais vous venez d'expliquer à juste titre que la création de lignes de covoiturage express peuvent en effet parfois se révéler

qui vote contre qui s'abstient il est adopté nous continuons par l'amendement dix huit c'est m erix je vous en prie cher collègue oui madame la présidente monsieur le ministre chers collègues le terme c'est d'abord cela vient d'être rappelé tout à l'heure le résultat de la coopération entre la région et la métropole la région, responsable de la planification des mobilités, la région, aussi compétente pour décider du nombre de trains et de car express La métropole, autorité organisatrice des mobilités, de l'intercommunalité centre. c'est elle qui anime l'action dans le périmètre, qui est principalement à l'œuvre pour que les conditions d'intermodalité d'urbanisme ete aussi active cette grande affaire, alors euh il s'agit bien il faut garder ce caractère coopératif coopératif au terme, c'est ce qu'avait prévu l'assemblée nationale en prévoyant que la demande de statut, l'attribution du statut de E R. M. soit une demande conjointe de la région et de l'autorité organisatrice de mobilité. Il serait étrange que ce soit le Sénat qui éclipse le territoire, Merci, cher collègue M. le rapporteur, l'avis de la commission. central aux régions dans la labellisation du Er M. Compte tenu de leur rôle de chef de file en de matière de mobilité, j'ajoute que les O M que les O M seront évidemment associées à l'ensemble du processus puisqu'elles seront partie prenante à la fois de la concertation préalable prévue à l'article 1ᵉʳ, Elles seront également à l'initiative aux côtés des régions pour permettre à la G P d'intervenir, le cas échéant dans l'élaboration et la maîtrise d'ouvrage d'un sermon il me semble que nous avons trouvé là un équilibre qui est satisfaisant. Pour ce qui est de la labellisation, gardons nous encore de complexifier davantage ce processus? Je vous propose de retirer votre amendement, sinon je donnerai un avis défavorable, merci M. le rapporteur, M. le ministre. Oui, Mᵐᵉ la Présidente, j'émettrai le même avis. je pense que, d'une part, il faut être un pilote. Le pilote, ce sera dans la plupart des cass des régions, évidemment en lien avec les métropoles et d'autres autorités organisatrices, si besoin, on couvre l'essentiel et il faut que ce chef de file si je puis le dire soit bien clair ensuite il existe des outils de coopération feront qui se fera par ailleurs naturellement je le pense mais si besoin, il y a le contrat opérationnel de mobilité qui est prévu par la Lomi existe et qui permet de réunir les différentes M. Donc, je suis comme le rapporteur d'avis qu'on n'alourdisse pas trop et qu'on trop et qu'on ne formalise pas excessivement la procédure. M. le Ministre, je mets aux voix cet amendement avec deux avis défavorables de la Commission et du Gouvernement, qui votent pour

nous l'avons pointé, c'est toutes les limites de ce texte il n'y a pas d'engagement clair sur les moyens financiers et budgétaires alloués par l'état pour permettre la création des services express on a bien entendu évidemment, la parole de M.. le ministre qui s'engage mais donnés mal quand c'est dans le texte en tout cas c'est mieux il y eu des améliorations en commission, c'est vrai et un plan de financement devra être établi avec une participation de l'état en lien avec les collectivités. Cette participation devrait selon nous tenir compte des différences des ressources entre les régions de France et, plus largement, entre les collectivités concernées par les Er Le soutien à la transition et à la mobilité doit pouvoir se faire en distinguant les besoins plutôt qu'en renvoyant les collectivités face à des réalités budgétaires parfois difficiles et toujours contrainte. Il y a région les régions, collectivités et collective. Je pense que l'on vit pas tous la même chose euh sur le territoire français il faut savoir en prendre compte

texte. Chers collègues, l'avis de la commission sur cet amendement. prenant d'ores et déjà en compte les capacités de financement de chacune des régions, les P E R qui sont par ailleurs en cours de négociation permettent aux régions d'exprimer permettent aux régions d'exprimer leurs besoins et attentes et c'est également dans cette démarche que le conseil d'orientation des infrastructures dans dans lequel je siège à travailler. Donc, Donc, je vous demande un retrait, sinon un avis défavorable. M. le rapporteur, le ministre, oui, Mᵐᵉ la Présidente, un avis défavorable également, je crois qu'il faut pas qu'on mélange les outils. La La péréquation, c'est essentielle mais on a déjà un certain nombre d'outils, notamment à travers la D G F et sa part consacrée à la notation de péréquation les Serbes eux mêmes ce n'est pas en soi un outil de péréquation, même s'ils luttent par nature contre les inégalités territoriales et évidemment dans la discussion qui se fera au cas par cas l'état tiendra compte des capacités contributives des différentes autorités organisatrices, mais je préfère qu'on ne mélange pas nos outils budgétaires de relations entre États et collectivités, il ne s'agit pas ici de créer une forme de dotation interne, de péréquation formalisée et par avance au sein des Merci

la présidente là on reparle d'interopérabilité et de bill éthique comme j'ai pu le dire tout à l'heure quand on avait des amendements en discussion commune qui ont été adoptés nous avions fait le choix d'intégrer la problématique de l'interopérabilité au niveau de l'alinéa 12, c'est l'alinéa par arrêté ministériel la création du Cer M, et donc on avait proposé la phrase à cet endroit que s'est arrêté On permet aussi d'étudier les conditions garantissant l'interopérabilité des services d'information des voyageurs et de bie éthique.

c'est le seul moyen de citer les habitants des agglomérations concernées à faire le choix de laisser leur voiture en fluidifiant des transports en commun. le conseils d'orientation des infrastructures donne une définition, un objectif simple, une fréquence à l'heure de pointe inférieure à 20 min et 1 h de creuse inférieure à 60 min. C'est une fourchette assez large mais qui a le mérite de déterminer un objectif, votre amendement nee donnee pas d'objectifs chiffrés mais plutôt une orientation générale qui permet de laisser une liberté d'appréciation aux collectivités dont ce sera la compétence. c'est dans ce sens qu'il faut faire progresser ce texte. Nous craignons dans le cas contraire et j'espère me tromper de créer un simple label avec une proposition loin, un peu marketing. Mais voilà, je l'essentiel de l'intervention est là. Cher collègue, avis de la commission

principe que le contrat opérationnel de mobilité et et c'est là où on va définir les objectifs les modalités d'action des différentes autorités organisatrices de mobilité en outre je qu'il est important de laisser la souplesse à la région, aux différentes O M dans la conclusion de leurs contrats opérationnels de mobilité, mais je pense qu'elles le tendront toutes à aller v. les objectifs que vous avez fixés et rappelés, et qui apporteront une réelle amélioration de la qualité des services, et pas exclusivement une labellisation, qui n'aura pas d'effet positif sur les usagers, avis défavorable s'il n'y a pas de retrait. M. le Ministre, avis du Gouvernement sur cet amendement numéro deux Même avis défavorable, Mᵐᵉ la Présidente, puis pour en dire un mot, M. le sénateur Barros, il s'agit là aussi de préciser de fait, à travers votre amendement le contenu des contrats opérationnels mobilité, je pense que c'est un outil qui fonctionne bien, qui doit être fonctionné encore un peu davantage et être mieux approprié, si je puis le dire ainsi. Mais Mais préciser ou complexifier, d'une certaine façon, davantage son contenu par rapport à ce qu'est prévu dans la Lom me paraîtrait ici, là aussi, un peu superflu ou excessif, donc je pense que cet outil existe et que c'est ainsi qu'il faut utiliser pour répondre. bien. Je mets aux voix cet amendement avec deux avis défavorables de la commission et du Gouvernement, qui vote pour

de nos déplacements et de la mobilité en moyenne les français font trois trajets par jour pour une durée d'environ une heure lorsqu'ils font ces trajets en voiture avec un véhicule thermique il contribue thermique deux du secteur des transports ce qui est quand même pas mal les études montrent qu'il y a pourtant des rapports modaux possibles c'est à dire des alternatives à la voiture moins polluantes et qu'il nous faut donc soutenir la voiture est utilisée pour de petits trajets des trajets courts de moins de kilomètres alors que trente pour cent des français les font à pied cinquante deux pour cent prennent leur voiture c'est ce genre de pratiques qu'il faut également inciter à changer notamment en renvoyant les aménagements piétons et cyclables il faut aussi reconnaître que nous allons plus loin depuis que la voiture est démocratisée et nous avons vu naître des zones commerciales des zones industrielles en dehors des villes et noushabadi de nos lieux de travail. Il y a donc aussi un enjeu de redynamiser les villes et permettre une densité de logements avec des prix accessibles aux abords des gares et de développer ces services, les commerces et les emplois de proximité, pour accompagner l'ensemble de ces démarches nous proposons qu'il y ait un objectif clair de report modal pour que la qualification de E R M soit associées à une baisse de l'utilisation de la voiture au bénéfice de modes de transport moins émetteurs de O deux et donc plus respectueux de l'environnement et de la qualité de l'air. chers collègues, l'avis de la commission sur ce Mᵐᵉ Mᵐᵉ la Présidente Storrs, pour les mêmes raisons que l'amendement précédent, je vais donner un avis défavorable, à la fois, le fait que le contrat opérationnel de mobilité a déjà pour objectif de déterminer entre les O M et entre les O M et la volonté de laisser aux O M décider librement du contenu précis de leur contrat, même si on partage également le constat que vous avez pu faire sur beaucoup de points, avis défavorable.

Le report modal ou ou finalement la le la possibilité pour le transport collectif de gagner sur la voiture individuelle c'est quand même prévu dans l'article 1ᵉʳ puisqu'il y a la possibilité qui est écrite de, pour les collectivités, de d'aller prendre notamment des sites propres, des voies réservées pour les transports collectifs et d'inciter cette pratique. il y a donc quand même cette volonté d'aller grignoter sur la voiture individuelle sur l'auto soliste pour développer les transports collectifs

participe activement à la rédaction de schémas de planification ayant trait au volet mobilité, il faut leur donner du sens. C'est notamment le cas des schémas de cohérence et d'organisation territoriale. Les scots bien sûr les plans locaux d'urbanisme ou encore au niveau régional le pour cela Le présent amendement vise donc à valoriser le travail effectué et à souligner le caractère essentiel des contrats opérationnels de mobilité pour le bon fonctionnement et la déclinaison des projets de E M et leur consultation par les élus locaux concernés et en 1ᵉʳ lieu les maires en ce sens. La co construction du contrat opérationnel de mobilité en coordination avec les schémas de planification communaux, régionaux et départementaux métropolitain peut faciliter l'obtention du statut de Ser Mp prévu par cet alinéa. Voilà donc le sens de cet amendement, cher collègue, l'avis de la commission. Mᵐᵉ la Présidente, sénateur gilet, la cohérence entre le contrat opérationnel de mobilité et les schémas élaborés par les différents échelons de collectivité est en effet nécessaire. Pour autant, cett amendement à notre sens est d'ores et déjà par l'article cinq d de ce texte qui étant au serbe la possibilité de recourir à la procédure intégrée pour mettre en compatibilité les différents documents d'urbanisme et puis vous le verrez lors de l'amendement trente et un de votre collègue jacquin la commission a émis un avis favorable à cet et il va vous satisfaire par rapport aux objectifs qui étaient ceux de cet amendement donc je vous propose de retirer cet amendement auquel cas je serai dans l'obligation de donner un avis défavorable M. le rapporteur, M. le ministre. Oui, Mᵐᵉ la Présidente, je partage aussi l'analyse du rapporteur Cet amendement sera satisfait, donc je propose d'en assurer le retrait, sinon je donnerai un avis défavorable, Merci, M., Gilet, je vous en prie. donc, en fonction de ces éléments, je vais le retirer, mais je voudrais quand même préciser qu'il faudrait que inscrire euh dans les scots et dans les l e i euh justement, l'intégration de ces volants de ces volants mobilités en termes de complémentarité avec les Ser Mes c'est à dire qu'il y a des clauses de révision à un moment donné on tu peux très bien annexer dans un 1ᵉʳ temps et puis ensuite dans le cadre des clauses de révision, faire en sorte que les L. E. I. les scots s'adaptent donc à ces nouvelles modalités ce qui permettraient

madame la présidente je v vous proposer s'il vous plaît un très bon amendement un amendement qui porte sur un sujet majeur celui de la sûreté dans les transports d'une nouvelle offre grâce aux services express régionaux métropolitain devra s'accompagner d'une réflexion sur cette problématique en amont Cet amendement vise à ce que, dans l'ee où les départements accueillant un R M le représentant de l'état dans le département réunissent les parties prenantes afin d'élaborer un contrat d'objectif départemental

Quel est votre avis? Oui, euh. J'y suis favorable, je pense qu'on est dans deux débats qui s'entrecroisent, évidemment, l'organisation d'une offre de transport supplémentaire c'est l'objet de la proposition de loi et des Ser Mes et puis la question plus large évidemment est évidemment importante encore davantage, malheureusement aujourd'hui, de la sûreté pour les usagers si on peut trouver à cette occasion une flexibilité supplémentaire qui permet d'inclure davantage de départements et de collectivités dans ces contrats je pense que c'est une bonne de le faire et cela n'épuise pas évidemment le sujet de la sécurité, de la sûreté dans les transports, je sais M. le rapporteur votre engagement sur ce sujet, nous aurons l'occasion d'en rediscuter C'est donc une étape utile que vous proposez à travers cet amendement je le redis, j'y suis favorable

Pour répondre réellement à cette ambition, il convient de s'assurer que les besoins de tous les citoyens et de tous les ont été correctement identifiés pour cela le contrat opérationnel des mobilités qui doit décliner les réponses à ces besoins en termes d'offre de transport et de complémentarité entre les territoires, gagnera en pertinence et en légitimité, s'il se fonde sur une participation citoyenne préalable à la conclusion du contrat opérationnel de mobilité Cet amendement vise donc à ancrer les décisions du contrat opérationnel dans une légitimité démocratique et une acceptation solide des citoyens et de leurs représentants. Le dispositif d'association vise également à renforcer la portée du contrat opérationnel en exposant par les différents éléments du dossier à une politique de transport pour toutes et tous, au service des territoires. Voilà le sens de cet amendement.

des citoyens et notamment des futurs usagers des desserts mais est évidemment une étape clé leur déploiement et pour qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions pour autant la Commission est défavorable, au moins pour trois raisons il existe déjà des instances permettant de les associer aux choix opérés en matières de mobilité. je pense notamment aux comités des partenaires,

des habitants également des consultations et études préalables au projet de ce type. Donc, on pense que, avec cet amendement, on va un petit peu plus complexifier les choses et c'est la raison pour laquelle on vous demande un retrait ou un avis défavorable. Merci M. le rapporteur, avis du Gouvernement. Oui, même avis, Mᵐᵉ la Présidente, avec des arguments similaires là aussi, faisons confiance à l'organisation locale, aux collectivités qui vont assurer ce débat et ces modalités peutêtre qui différeront légèrement d'une collectivité et d'un projet et d'un projet à l'autre, de participation citoyenne et comme l'a rappelé le rapporteur il yy a en effet d'autres instances qui sont notamment dédiées à consultation à ce travail plus large c'est notamment le comité des partenaires. Donc, je vous demanderai le retrait à défaut je donnerai un avis défavorable également.

de faire participer d'expliquer sur les questions de mobilité, on sort d'une campagne électorale et sénatoriale, Moi, il me semble qu'il n'y a pas un endroit où je sois allé, il n'y a pas une commune, il n'y a pas une métropole, justement, de ces questions de mobilité justement de ces questions de mobilité et donc un vrai besoin en tout cas à la fois d'écoute de lien avec les citoyennes et avec les citoyens alors je ne sais pas si c'est forcément le bon vecteur via cet amendement mais en tout cas, moi, il me paraît particulièrement intéressant d'appuyer sur sur cette participation citoyenne, notamment avec les contrats opérationnels, de de mobilité et que cela soit construit avec les citoyens et c'est vrai que vous parlez des des des L d des comités, de partenaires. Il me semble que ce n'est pas tout à fait le même dispositif L là, on est sur la construction justement d'un service express régional métropolitain on doit associer et l'associer à toutes les étapes l'ensemble des citoyens. Cher collègue, il n'y a plus d'explication de votre, je n'en vois plus. Je vais donc mettre aux voix cet amendement avec deux avis défavorables de la commission et du Gouvernement qui vote pour Qui vote contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté, amendement 14 M.. le Ministre, un amendement du Gouvernement. Oui, Mᵐᵉ la Présidente, M. le rapporteur, j'ai presque des à rendre à rendre cet esprit presque unanime, hein S, sur beaucoup de sujets, voire d'amendements, mais je me dois quand même de signaler ce point. Un amendement qui revient, en effet, sur les travaux conduits en commission. Une volonté partagée, c'est la question des péages et de la tarification du réseau et j'ai lancé cela a été évoqué par plusieurs d'entre vous pour la 1ʳᵉ fois. Je crois, avec Bruno Le Maire, une mission sur la tarification et le niveau des péages ferroviaires en France. De manière générale, j'ai quelques difficultés à faire une forme de catégorie spécifique pour les Serbes, même s'ils sont très importants, parce que il y aura forcément des entre croisements. Des E R, par exemple, qui vont faire partie des Serbes qui pourraient être mieux cadencés, plus nombreux, avec éventuellement quelques lignes nouvelles, vont parfois circuler en dehors du périmètre des termes eux mêmes et il n'y a pas tellement de raisons d'avoir une forme de tarification facilitée ou favorable dans le périmètre du sert mais de ne pas avoir ce même débat et cette même tarification. favorable si on doit la faire évoluer de manière plus globale pour des trains express régionaux qui se situeraient en dehors de ce périmètre. Donc je partage l'idée avoir une réflexion sur la tarification et sur le niveau des péages qui, en France, en effet, posent un certain nombre de difficultés. Nous avons lancé ce travail, mais je pense que l'articuler ou l'associer directement à la notion de Serbo serait un certain nombre de difficultés, c'est la raison d'être de cet amendement non pas pour me détourner de la préoccupation que l'on partage, mais pour assurer cette cohérence, je vous remercie. le ministre, M. le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur cet amendement du Gouvernement? lé à mon tour, M. le Ministre, tout se passait bien, vous l'avez dit jusqu'à présent je vais être dans l'obligation de donner un avis défavorable à votre amendement parce que c'est un sujet qui, vous le savez nous Nous mobilise particulièrement dans la commission

malheureusement le niveau des péages dans notre pays ferroviaire pénalise ceux qui veulent faire pluss de train et ceux qui veulent mettre en place le choc d'offre que l'on attend tous donc c'est la raison pour laquelle, tout en regardant avec beaucoup d'attention, la mission que vous avez lancée et le travail de de de l'i G F. Euh sur ce sujet. Euh, nous préférons conserver notre amendement, et il nous semble que on peut, à travers cet amendement, constituer un levier concret en faveur du renforcement de l'offre, en tout cas, nous l'espère ainsi, et je vous propose de donner un avis défavorable au à l'amendement du Gouvernement. Merci M. le rapporteur, alors j'ai plusieurs explications de votre M. Jacquin tout d'abord. Très succinctement, pour aller dans le sens du rapporteur, on a l'occasion là de porter le débat sur la tarification des péages en France, qui est un véritable problème ferroviaire puisque nous avons les péages parmi les chers en Europe et qu'actuellement parler de choc d'offres avec cette tarification des péages n'est pas une bonne occasion le rapporteur nous a donc permis d'introduire la possibilité de réfléchir à la tarification de ces péages. Je pense qu'il faut en profiter pour améliorer la réflexion sur ce sujet important et permettre ainsi un développement du ferroviaire. Enfin, je tiens à dire que Il y a un piège derrière cess histoires de tarification il faut pouvoir couvrir le coût complet du gestionnaire d'infrastructures N C F réseau et dans bien des pays où les péages sont moins chers, il y a des subventions d'équilibre qui sont données, donc c'est la précision que je voulais apporter, on n'a rien sans rien et il faudra bien couvrir, les coûts complets et cela ne peut se traiter, au seul coût marginal d'exploitation je vous remercie remercie cher collègue monsieur fernie que vous vouliez également intervenir pour une explication de votre je vous en prie que euh ça vient de dire les péages parmi les plus élevés d'europe et un contrat de performance n c f réseau qui mise sur une augmentation de vingt huit de ces péages parmi les plus élevés autrement dit l'effort pour la régénération pour la modernisation il est assis sur cette hausse des péages alors au moment où d'activer, d'aider, d'accompagner l'intensification de nos circulations E R sur les bassins de mobilité de nos métropoles, au moment où on cherche à optimiser l'usage de ces infrastructures. Je crois qu'il faut que le Sénat donne le signal politique qu'il faut cesser avec cette logique contradictoire mon cher collègue, M. le ministre. Simplement, pour être très clair, la question des péages est une question importante on doit la traiter, je pense qu'elle dépasse la question des Serbes mais je prends si vous me permettez cette expression juridiquement incorrecte M.. le rapporteur travaux de la Commission comme une cours des travaux de la Commission comme une forme d'appel à faire mieux sur la question des péages ou à rouvrir cette question à travers le sujet des S R M pour répondre aussi à M. Fernicle

pourraient être au total maintenu voire améliorée parce que ce que je ne veux pas faire c'est baisser les ressources au moment où doit justement les augmenter de N c f réseau puisque N c f réseau puisqu'on a tous dit depuis le début de cette discussion que que la priorité des priorités c'était d'investir dans la régénération et la modernisation durée ferroviaire c'est pour cela que la mission doit éclairer ces options. Elle sera de toute façon évidemment rendue publique et présentée au Sénat comme à l'assemblée nationale. M. le Ministre, je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement avec je vous rappelle un avis défavorable de la commission qui est pour cet amendement

gillet madame la présidente vous l'avez compris nous estimons qu'il n'est guère pertinent de limiter l'ambition de la mise en place de e m en ne prévoyant que dix au contraire nous proposons donc en cohérence nos amendements précédents d'élargir donc et de basculer dans un nouveau modèle fondé sur des services express de mobilité généralisé à l'ensemble des bassins de mobilité en deux mille dix neuf et constituant depuis un nouvel espace de référence en matière de mobilité la lomm a en effet chargé la région en tant que chef de file d'organiser les modalités de l'action commune des oem sur les différentes formes de mobilité d'intermodalité les desserts la création l'aménagement le fonctionnement des pôles d'échanges multimodaux l'aide à la conception, la mise en place d'infrastructures de transport, de services, de mobilité, Pour les autorités, que ces actions s'exercent à l'échelle des bassins de mobilités, considérés comme l'échelle représentative. de la mobilité au quotidien, la loi prévoit aussi qu'il revient aux régions de définir et de délimiter, en concertation notamment avec les o m les syndicats mixtes de transport et les départements ces bassins de mobilité la proposition de loi que nous examinons vise à déployer des services express régionaux de mobilité C comme devant correspondre à des services quotidiens de mobilité de haute qualité, intégrant une offre interne et multimodale qui doit irriguer donc les territoires. Il s'agit de créer un véritable choc d'offres de mobilité au quotidien mais pas seulement ferroviaire, capables de rayonner autour des pôles d'attractivité que sont les métropoles et d'irriguer l'ensemble du bassin de mobilité. L'échelle du bassin de mobilité devrait précisément permettre de mailler le territoire en service collectif, publii de mobilité. nécessairement nécessaire aux déplacements du quotidien des populations, c'est donc le sens de cet amendement en termes d'élargissement à l'échelle des bassins de mobilité. Chers Chers collègues, l'avis de la Commission sur cet amendement, Mᵐᵉ la Présidente, Slater Gilets nous comprenons une nouvelle fois votre démarche d'élargissement des serres au delà des centres urbains et périurbains mais la Commission a émis un avis défavorable pour deux raisons à la fois. La référence au bassin de mobilité n'est sans doute pas la plus opérante pour définir où déployer il n'est peut être pas pertinent pour chacun des bassins de mobilité de créer un terme, il faut savoir se donner des des objectifs qui soient peut être atteignables déjà la réalisation d'i cerfs d'ici 10 ans est ambitieuse celle de créer des serma bassin de mobilité sans distinction. Heuh peut être utile mais semble peu réaliste. merci M. le rapporteur. avis du gouvernement. euh même avis, M. le sénateur Gilet que celui exprimé par le rapporteur. Deux choses la notion de la notion de bassin de mobilité est intéressante mais elle ne correspond pas ou ne se confond pas je pense qu'elle ne doit pas se confondre exactement avec les services express régionaux métropolitains comme l'a dit M. le rapporteur il peut y avoir des bassins de mobilité des bassins de mobilité où il n'y aura pas ou pas tout de suite le service express régional métropolitain et inversement des termes y compris dans les projets qui sont déjà envisagés qui peuvent couvrir cinq à dix bassins de mobilité puisque dix bassins de mobilité puisque je crois qu'il y en a aujourd'hui plus de deux cents qui sont recensés en france en revanche pour répondre sur le fond à la préoccupation que vous exprimez la liste n'est pas arrêtée c'est à dire qu'il y a des travaux qui ont été faits en deux mille vingt par s n c f réseau quii ont servi de fondement au rapport du conseil d'orientation des infrastructures cela fait je simplifie entre dix et quinze métropoles qui pourraient rentrer dans une première vague évidemment le souhait c'est que ensuite il puisse y avoir d'autres projets qui soient présentés et qu'on avance même si comme l'a rappelé le rapporteur soyons d'abord d'abord mais crédibles et réalistes. il faut réussir une 1ʳᵉ vague de projets on peut en lancer d'autres mais tout cela prendra un peu de temps mais en tout cas, je veux être rassurant et clair il n'y a pas une liste fermée de service Express Région métropolitain qui sera définitivement arrêtée dans quelques mois euh pour solde de tout compte en quelque sorte. sorte. M. le Ministre, je vais donc mettre aux voix cett amendement qui a reçu deux avis défavorables de la Commission et du Gouvernement qui votent pour, qui votent contre. qui s'abstient, il n'est pas adopté. je vais donc mettre aux voix l'article premier qui vote pour l'article

gillet madame la présidente il convient de s'assurer dans le c le cadre d'un service express régional métropolitain que le contrat opérationnel des mobilités prévoit bien des moyens d'accès aux services à l'ensemble des populations du territoire, y compris celles qui seront les plus éloignées des gares et des stations avec une attention particulière pour les populations qui peuvent rencontrer spécifiques. Cette disposition vise à mettre en œuvre une vision globale, anticipée et coordonnée de cette problématique d'accès pour le plus grand nombre au service express métropolitain en complémentent notamment de la disposition de l'article deux qui prévoit que les collectivités locales ou leurs groupements

Mᵐᵉ la Présidente, le sénateur Gilet cet amendement est déjà satisfait par le droit existant. Le code des transports prévoit déjà que le contrat opérationnel de mobilité porte notamment sur les différentes formes de mobilité et l'intermodalité et la création des des Pmes la Commission partage votre souci que les serves bénéficient aux territoires les moins denses, là les moins denses. Là encore, il est déjà prévu que le contrat porte sur la création l'aménagement le fonctionnement des des aires de mobilité, notamment en milieu rural et qui comprennent les dispositions spécifiques concernant l'accueil de tous les publics et la cohésion sociale. Une grande souplesse quant au contenu du contrat doit être laissé aux acteurs locaux. Je vous propose un avis défavorable merci monsieur le rapporteur l'avis du gouvernement

sont un bon dispositif du quotidien il conviendrait de les étendre cet amendement visait à faire en sorte qu'au delà de la métropole dans les territoires périurbains qui sont en aval soit parfaitement prises en compte c'était cela et c'était donner une garantie que, comme vous nous l'avez dit, la métropole nee va pas s'occuper que du cœur s'occuper que du cœur des métropoles. mais verra bien comment desservir les habitants qui sont les plus éloignés du périmètre du cœur de cette métropole. Donc, nous maintenons cet amendement merci cher collègue bien donc je mets aux voix cet amendement avec deux avis défavorables de la commission et du gouvernement qui votent pour qui vote contre

des employeurs et des usagers, ce qui est évidemment une très bonne chose mais au regard de l'ampleur des projets dont nous parlons. les services express régionaux, et des et des attentes très fortes, en particulier dans le domaine du ferroviaire, il nous semble absolument indispensable d'élargir la composition de ces comités, des partenaires nous l'avons redit euh. Les montants de dépenses publiques sont quand même considérables en ce qui concerne l'ensemble de nos concitoyens. Les attentes en matière de services de de mobilité sont là aussi très prégnantes et cela concerne donc très largement nos concitoyennes et nos concitoyens et pour toutes ces raisons là, il nous semble donc essentiel d'élargir cette composition et de favoriser une meilleure reconnaissance des corps intermédiaires ceux là même qu'ils sont parfois trop souvent en tout cas mépriser ou oublier en particulier les organisations syndicales et les acteurs associatifs. Nous vous proposons d'ajouter ces deux catégories d'acteurs à la composition des comités de partenaires. Je vous remerci, cher collègue, ami de la Commission. Mᵐᵉ la Présidente, Senator Usa, le code des transports prévoit que le comité des partenaires comprend a minima des représentants des employeurs et des associations. d'usagers ou d'habitants ainsi que des habitants tir au sort. Il revient ainsi aux autorités organisatrices de la mobilité de fixer leurs Il est donc d'ores et déjà possible d'intégrer des représentants D d'association ou encore des organisations syndicales, de salariés. J'ai pour mémoire que c'était le cas en région Provence halet d'azur où nous avions toutes les organisations syndicales qui étaient représentées. Voilà donc, je pense qu'on va pas le mettre dans la loi, qu'il faut laisser la main au Zao pour ne pas rigidifier les compositions des comités de partenaires, mais tous les Os auront, je l'espère, et je n'en doute pas un instant la bonne idée de de prévoir une concertation la plus large possible avec notamment les organisations syndicales de qualité, que nous avons dans notre pays,

J'ai bien entendu la position de M.. le rapporteur, pas plus que cela, et on peut partager un certain nombre de points, notamment sur la capacité des acteurs locaux, des élus, à prendre en compte ces réalités là. Pour autant, là. Pour autant, la loi et les mots ont un sens et c'est vrai qu'aujourd'hui cette approche de notre point de vue trop restrictif mentionné uniquement les employeurs. nous Nous nous semble regrettable dans un moment où, a fortiori, nous avons besoin d'un dialogue social renforcé et nous avons, de notre point de vue, aussi besoin d'associer, dans le cadre de ces projets structurants, celles et ceux qui vont contribuer très largement à leur production, à leur mise en œuvre, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons a minima, donc, de rectifier cet amendement et de proposer simplement l'élargissement des comités de partenaires, aux seules organisations syndicales, mais parce qu'encore une fois, cela a un sens. et les employeurs et les organisations syndicales de pouvoir les prendre en compte dans une logique dans une logique paritaire. Donc j'espère que M. le rapporteur vous serez sensible à cette évolution. Je vous remercie. Merci, cher collègue, plus d'explication de vote? Non, je mets donc aux voix cet amendement. M.. le rapporteur, sur la demande présente de mon président de la commission. Et par rapport aux arguments qui ont été euh, euh qui ont été données et par rapport du Gouvernement, même sii je pense que les partenaires l'auraient fait euh d'même enfin, les autorités l'auraient fait de même, je vous propose qu'on donne un avis favorable ou en tout cas un avis de sagesse, à cet amendement, un avis de sagesse. d'accord bien, alors, cet amendement a recueilli deux avis de sagesse de la Commission et du gouvernement qui votent pour qui vote contre alors qui s'abstient il est adopté

ont donc des interactions indispensable avec les territoires métropolitains et elle devrait donc être être également intégrée par représentation la gouvernance des services express métropolitains et donc cet amendement vise Àde à la société des grands projets et à la société nationale ne Pour une meilleure prise en compte justement de la réalité de ces territoires la composition du conseil de surveillance de la société du Grand Paris devenant société des grands projets doit nécessairement être modifié pour tenir compte de l'évolution de son périmètre d'action. Cette disposition appellera donc une modification du décret précité relatif à la Société du Grand Paris. conséquent, taille aujourd'hui très restreinte du conseil d'administration de la n c f douze membres permett d'envisager aussi une telle extension tout en maintenant l'effectif du conseil dans les normes des grandes sociétés quinze ou dix huit membres voilà donc le sens de cet amendement merci cher collègue avis de la commission madame la présidente sénateur gilet je comprends parfaitement votre volonté d'adapter la la gouvernance de la g

concernant le cas de la N C F Il nee semble pas. Idoine de faire entrer dans son conseil de direction ou son conseil de surveillance des représentants surveillance des représentants des communes ou des intercommunalités de moins de 10 habitants, il serait en effet peu justifié de choisir ses représentants plutôt que d'autres, pourquoi pas des représentants des Conseils régionaux par exemple outre le choix laissé dans vostre amendement entre le conseil d'administration celui du conseil de surveillance me semble être source d'un manque de clarté ou de lisibilité de la loi, donc je donnerais un avis défavorable. Sieur le rapporteur, M. le Ministre, avis du Gouvernement? Oui, Mᵐᵉ la Présidente, le même avis que M. le rapporteur, avec les mêmes arguments. je mets au voix cet amendement qui a recueilli deux avis défavorables de la commission et du gouvernement qui vote pour

dont la composition doit comprendre a minima le conseil régional le p c i ou l'agglomération centrale de l'étoile concernée ce i p doit s'assurer les projets de R M et leur impact direct comme indirect, s'inscrivent en cohérence avec les schémas régionaux et locaux de programmation

des schémas de programmation territoriale et est donc eston pertinent que tout au long de la réalisation les maîtres d'ouvrage veillent au respect de ces schémas confier cette mission aux groupements d'intérêts publics les réunissant est opportun puisque ces groupements à un rôle de coordination de l'action des maîtres d'ouvrage donc je donne un avis favorable bien sûr et sous amender un sous amendement de coordination numéro soixante deux merci monsieur le rapporteur monsieur le ministre sur sous amendement ensuite l'amendement s'il vous plaît oui si vous me permettez de répondre globalement tel que sous amendé je peux donner un avis favorable à l'ensemble qui serait ainsi ajusté monsieur le ministre il y a deux avis favorables de la commission et du gouvernement sur cet amendement sous amendé je mets aux voix le sous amendement pardonnez moi qui vote pour le sous amendement qui est un sous amendement de coordination il est adopté donc qui vote qui s'abstient il est adopté et l'amendement qui vote pour. qui votre compte qui s'abstient, il est adopté bien. Je vous remercie. Je mets aux voix l'article un bis ainsi sous abandon qui votre pour

relevant du réseau de transport publics du grand Paris ou dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée, il ne serait pas cohérent que la G p nee bénéficie pas de ces exemptions également pour la réalisation des infrastructures déclarées d'utilité publique des services express régionaux métropolitains en île de France, alors même que le statut de ces services relève d'un arrêté du ministre chargé des transports sur la base d'une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes de pour l'organisation de la mobilité. C'est pourquoi cet amendement propose de compléter la modification apportée sur ce point, en visant également le cas où la maîtrise d'ouvrage d'un serme est confiée à la S.

conjointement par les ministres en charge de l'urbanisme et du budget la loi de juin deux mille dix relative au grand paris prévoit l'exercice d'une mission en matière d'aménagement et de construction celle ci similaire à celle des établissements publics d'aménagement étaient initialement articulés autour des contrats de développement territorial dont le champ est celui du grand paris il est par ailleurs considéré que la g p peut intervenir sur le territoire des communes non signataires en respectant certaines conditions les opérations ne peuvent être réalisées que dans un rayon de six cents mètres autour des gares du réseau de transports publics du grand paris et d'égards des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage lui a été confiée ds lors que la maîtrise d'ouvrage des gares des infrastructures des Serm pourrait être confiée à la G p. Cette disposition pourrait être trouvée à s'appliquer en dehors du territoire francilien.

au droit de priorité pour les projets e m et bienvenue et permett un parallélisme des formes avec les droits accordés à la g p dans le cadre du grand paris express donc avis favorable pour celui là je le trouve à la confusion au processus d'autorisation de la g p pour intervenir dans le cadre du déploiement des serbes les opérations d'aménagement et de construction de Saa maîtrise d'ouvrage en matière de E qui plus est par arrêté des ministres du Budget et de l'urbanisme alors même que l'autorisation même que l'autorisation d'intervention de la gp en maîtrise d'ouvrage relève d'un arrêté du ministre des transports et ne me semble pas opportun c'est la raison pour laquelle je donnerais un avis défavorable pour le

bien je vais mettre aux voix s'il n'y a pas d'explication de vote l'amendement cinquante quatre présenté par madame avez avec deux avis favorables de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté l'amendement cinquante trois qui lui a reçu un avis défavorable de la commission un avis favorable du gouvernement qui est pour

en commun et sont les 1ʳᵉˢ concernées par ces projets. Elles disposent ainsi d'une connaissance fine des enjeux pour les territoires au regard notamment de leur implication dans les contrats opérationnels de mobilité ainsi que le présent amendement vise à s'assurer que les collectivités soient impliquées dans les différentes étapes d'élaboration des projets de E R N, à savoir l'étude des propositions et le choix des maîtres d'ouvrage. Je précise que, dans la rédaction, au niveau de l'amendement, on parle bien d'insérer les mots et, le cas échéant, des collectivités territoriales concernées. Donc c'est un amende, merci, cher collègue, Merci, cher collègue, avis de la commission sur cet amendement. par décision du ministre à la demande de la région ou des Om compétentes satisfaisant le risque de multiplier ainsi les parties prenantes et de ralentir considérablement les projets j'accédais nées ont évidemment évidemment vocation à être consultées en amont pour les déploiements des Serbes. Donc, c'est la raison pour laquelle je confirme l'avis défavorable. M.. le Rapporteur, avis du Gouvernement, s'il vous plaît, oui, j'aurais le même avis, Mᵐᵉ la Présidente, parce que je pense que l'équilibre, là aussi, est déjà trouvé et je rappelle que l'intervention de la G P sera de toute façon strictement conditionnée à la demande et à la coordination préalable entre les collectivités concernées

qui est contre qui s'abstient il est adopté excusez moi je continuons monsieur tabar monsieur le rapporteur au nom de la commission l'amendement madame la présidente est un amendement rédactionnel quii lève une possible ambiguïté entre les notions de titres de créance émis par la g p et les emprunts bancaires qu'elle contracte l'avis du gouvernement surement de la commission favorable avis favorable sur l'amendement de la commission qui est pour

treize je suis économe en amendement madame la présidente mais celui important puisqu'il consiste à augmenter en portant à trente neuf milliards d'euros excusez du peu le montant maximum de l'encours en principal des emprunts contractés par la société du grand paris il s'agit de mettre en cohérence les moyens et la capacité d'intervention de la société du grand paris avec les exigences que nous portons pour elles notamment avec les investissements en île de France mais aussi ceux qui seront réalisés dans le cadre nous l'espérons de cette proposition de loi, c'est un amendement important pour assurer les moyens d'intervention de la Cité du Grand Paris sans que cela, je souhaite rassurer le Sénat à cet égard ne remet en cause le modèle financier de la société du Grand Paris. Nii l'horizon qui reste raisonnable et acceptable du remboursement de sa dette Bien évidemment, je crois que c'est un amendement nécessaire et d'équilibre. M. le Ministre, l'avis de la commission sur l'amendement du Gouv sommes favorables à cet amendement, Mᵐᵉ la Présidente, avis favorable je mets aux voix l'amendement du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour

soient internalisées à la fois pour des raisons d'efficacité en disant le temps passé sur les appels d'offres des réunions de négociations. Et enfin, nous ici d'avoir eu le plus grand chantier d'europe avec le Grand Paris Express

pour accroître humains de la g p étant malheureusement limités je ne suis pas opposé par principe au recours au cas par cas des prestataires externes cela étant je connais l'attachement de notre assemblée à cette question en outre évaluer les moyens d'internalisation de certaines missions dans le cadre du rapport annuel peut être intéressant, on va émettre un avis de sagesse qu'on de sagesse qu'on dira bienveillante. Si M. le rapporteur, avis du Gouvernement. Je serai un tout petit peu moins bienveillant mais je voudrais l'expliquer parce que je voudrais préciser deux choses d'abord, l'objectif n'est pas d'externaliser des missions, c'est bien de d'utiliser les compétences développées pendant plusieurs années par la société du grand Paris qui est en fait un certain de prestataires externes mais avant tout sa substance Si je puis dire de compétence qui sinon d'ailleurs, serait aussi perdue puisque ses effectifs si on s'en tenait la mission française aurait décroître et ses compétences à retourner dans le secteur privé ou ailleurs je ne sais pas mais en tout cas, je pense qu'on en ferait bon usage en gardant cette société du grand Paris devenue société des grands projets. Il faut garder de la souplesse parce que même si cela doit rester raisonnable et je sais que le scénarii est particulièrement attentif et qu'il puisse avoir l'occasion de temps en temps d'avoir des prestataires extérieurs sans en abuser, pas plus qu'elle nee le fait aujourd'hui, mais c'est une flexibilité qui est importante donc je vous en demanderai le retrait, sinon j'émettrai un avis défavorable.

madame la présidente monsieur l'objet de cet amendement est bien d'ajouter au développement du réseau ferroviaire l'enjeu de l'électrification nous avons pris dans l'objet de l'amendement L'exemple du réseau. de Strasbourg Euh, qui est largement en retard sur cette électrification Mais il y a d'autres lignes en France. qui attendent aussi ces de modernisation? je pense en particulier à une ligne en Bretagne, donc nous souhaitons mettre l'accent dans la continuité des propos que nous avons déjà tenus sur la régénération et la modernisation et la modernisation du réseau en mettant en avant ce point qui a une dimension évidemment écologique écologique et également économique pour la performance de notre réseau. Je vous remercie,

six ah c'est monsieur isa madame la présidente monsieur le ministre chers collègues continuité avec l'amendement précédent il s'agit de remettre au parlement six mois après la promulgation de la présente loi un rapport présentant la stratégie et le schéma d'électrification des lignes ferroviaires Encore une fois. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de Strasbourg. l'exemple aussi d'une ligne en Bretagne, la ligne Quimper Brest, mais il y en a bien d'autres dans il y en a a bien d'autres donc ce rapport permettra de faire le point sur ce sujet. Chers collègues, avis de la commission. madame la présidente je vais donner un avis défavorable puisque vous l'avez dit dans votre exposé des des motifs chers collègues cette cet amendement est déjà satisfait votre votre amendement quarante cinq que nous venons d'adopter merci monsieur le rapporteur avis du gouvernement sur cet amendement oui même avis pour les mêmes raisons monsieur retire

tenir compte, c'est son expression pour la mise en œuvre des contrôles et des sanctions dans le cadre des F e de l'état d'avancement d'un Erm dans les territoires d'un Je ne pense pas que ça soit la vocation de ce texte d'affaiblir les F E car cette disposition, je l'ai dit tout à l'heure d'entrée serait sans doute utilisée comme un prétexte à l'immobilise dans la lutte contre la pollution de l'air d'origine automobile elle serait aussi je le crois bien une entorse à l'article quarante cinq qui est au périmètre de cette p p l car je ne lis rien j'ai bien regardé dans les éléments de ce périmètre qui permettent de légiférer aujourd'hui sur les f et si cet article n'est pas prescriptif c'est à dire qu'il ne légifère pas sur les F E s'il n'est qu'une vague préconisation, c'est qu'il est inutile et donc qu'il faut voter mon amendement de suppression.

des contrôles compte du rythme du déploiement. Je rappelle que, dans mon rapport, en juin dernier, adopté par la Commission, j'ai insisté sur ce besoin de synchroniser. la mise en œuvre des F E et le développement d'offres alternatives, cet amendement va donc dans ce sens. Sans pour autant freiner, bien sûr, le déploiement bien sûr, le déploiement des zones à faible émission C'est la raison pour laquelle je vais formuler un avis défavorable à votre amendement. M. le rapporteur Av du Gouvernement Mᵐᵉ la Présidente, alors j'entends les arguments de M. le rapporteur en réponse à la volonté de rétablissement de la rédaction de M. le sénateur Pernik. je serais plutôt favorable à ce qu'on garde la rédaction initiale est donc favorable à l'amendement de M. Fernie, même si j'entends qu'il y aura encore un peu de travail pour bien montrer ce qui était l'objet de l'amendement de Bis, qui n'était pas une volonté de Rev de revenir pardon de rouvrir un débat de principe sur les zones à faible émission comme vous l'avez précisé monsieur le rapporteur mais est donc favorable à cet amendement

Oui, c'est encore un amendement qui vise à rétablir un article de l'assemblée qui concerne là les niveaux sonores maximaux admissibles dans le cadre du développement des ser ms en effet le développement de ces offres multimodales pose un défi aussi en termes de nuisances sonores

si belles nuit alors qu'actuellement en france les niveaux c'est soixante jours et cinquante cinq nuits il est donc nécessaire de définir des mesures concernant les niveaux sonores liés au trafic de er ms qui soient plus adaptés en diminuant progressivement les niveaux c'est ce que préconise en demandant qu'on prévoit par décret la révision des niveaux maximaux admissibles de bruit ambiant d'une infrastructure ferroviaire nouvelle. Merci, cher collègue, l'avis de la commission sur cet amendement. Mᵐᵉ la présidente. Cher collègue Fénix, l'article deux bis que vous souhaitiez rétablir est déjà satisfait par le droit nous en avions parlé en commission et serait source de d'un manque de clarté et de lisibilité de la loi le code de l'environnement prévoit déjà que l'autorité réglementaire peut par décret en conseil d'état les prescriptions applicables aux infrastructures nouvelles créer un deuxième renvoi à un décret n'apportera rien de pluss si ce n'est de la confusion en outre si cet article aboutissait à créer une réglementation spécifique au serbe il ferait peser un risque sur leur développement or rien nee justifie qu'un train roulant sur un réseau labellisé R R M soit soumis à une réglementation plus stricte

un Transilien de France d'uniformité et de lisibilité de la loi plaide pour le maintien d'une réglementation unifiée. C'est pourquoi la Commission a émis un avis défavorable. Mᵐᵉ la Présidente, c'est un débat que nous avons eu à l'assemblée nationale pour renforcer si je puis dire renforcer si je puis dire à l'occasion des Serbes et leur mise en place le combat contre les nuisances sonores Euh, il y avait un équilibre qui avait été trouvé à l'issue du texte de l'assemblée nationale, ou partage, ou je comprends la préoccupation de rétablissement qu'exprime M. Fernie m'en remettrai, à la sagesse du Sénat. Merci, M. le ministre, il y a donc un avis défavorable de la commission et un avis du Gouvernement sur cet amendement 20 qui est pour qui est contre, qui s'abstient il n'est pas adopté l'article deux bis a reste donc supprimé je mets aux voix l'article deux bis b qui est qui qui est contre qui s'abstient il est adopté nous continuons par l'amendement vingt quatre présenté par m g madame la présidente l'article de bis introduit par les députés et imposant l'étude d'un scénario alternatif de lignes dites à vitesse intermédiaire lors de l'établissement d'un projet de ligne ferroviaire à grande supprimé en commission par l'adoption d'un amendement du rapporteur. Les auteurs de l'amendement souhaitent rétablir cet article, qui permet de soulever l'enjeu du financement de nos transports collectifs structurants de nos transports collectifs structurants en 1ᵉʳ lieu ferroviaire ainsi que la répartition financière de ces investissements. Il en résulte la nécessité de produire un choc d'offres de transport, est essentielle mais ne se fera pas sans la définition de priorités et la possibilité de fixer ces priorités de financement visant à développer les transports du quotidien et à permettre un report modal massif pour sortir de l'auto soliste, en particulier dans les territoires périurbains et ruraux. Ainsi, cet amendement propose de créer les conditions d'un choix budgétaire à la fois sur la création de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse mais également sur les projets en cours, face au manque de visibilité auquel sont confrontés les acteurs les collectivités organisatrices. Il faut souligner que dans le contexte, nous constatons tous une dégradation des ratios financiers des collectivités et plus particulièrement des régions, avec des durées euh de remboursement d'emprunt qui s'allongent aujourd'hui Cet amendement vise à créer donc une souplesse dans les choix pour pouvoir rediscuter effectivement des priorités en permettant de mettre en avant des vitesses inférieures et donc des investissements moindres pour pouvoir les supporter

qui déclinait bien je crois la cohérence du scénario de planification écologique du conseil d'infrastructures structures, amplifier les efforts pour les lignes à grande vitesse Yy est explicitement mentionné comme non prioritaire régénération, modernisation, commande centralisées du réseaux Tvo, les priorités impératives pour le ferroviaire, en ce sens, donner les éléments du choix du choix entre grande vitesse et vitesse intermédiaire, comparer les scénarios, ça donnerait une chance à cette priorité qui permettra d'améliorer les performances ferroviaires plus de trains plus de robustes exploitation plus de régularité je crois que l'expérience du serm strasbourgeois nous indique qu'il faut aller franchement dans ce sens

le mécanisme de financement des Ser mes proposé par ces deux amendements est inopérant d'éventuelles économies sur un projet par rapport à une autre version de ce projet nee sont en rien gain financier réellement disponible pour être investi dans les projets de R M. annexer le programme annuel d'investissement de N C F réseau à son contrat de performance comme le prévoit le texte de Commission devrait permettre de répondre à l'attention de cett amendement, qui est de soutenir nous l'avons bien compris les investissements en faveur des Ser Ms et des petites lignes, c'est C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements M.. le rapporteur, avis du Gouvernement. Mᵐᵉ la Présidente, il s'agit aussi de points qui aient fait l'objet de discussions et d'ajouts au cours de la discussion en hémicycle à l'assemblée nationale j'émettrai sur ces deux amendements un même avis de sagesse disons de sagesse bienveillante merci monsieur le ministre je vais donc mettre aux voix l'amendement vingt quatre qui a eu un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse bienveillante du ministre qui vote pour

qui s'abstient il n'est pas adopté nous continuons donc l'article deux bis est toujours supprimé nous passons à l'article trois avec un amendement trente sept présenté par monsieur oui oui pour évoquer les questions très importantes de sécurité ferroviaire dans l'article trois on prévoit que la g p ou sa filiale conclut une conventions avec N C F Réseau et les cas échéants sa filiale, Gare et Connexion, lorsque le ministre chargé des transports lui confie la maîtrise d'ouvrage pour une infrastructure ferroviaire nouvelle du réseau ferré national incluse dans un Er m dans le cadre de cette convention de gouvernance technique il convient à l'égard

les incidences du projet sur l'exploitation qui reviendra in fine à la N c f réseau, doivent également être précisément décrites afin de s'assurer qu'une fois le coût de réalisation couvert. on ne reporte pas de façon indirecte, une charge excessive de l'exploitation ainsi que cela a pu être par exemple constatée dans le passé en termes de projets de G V réalisés par des concessionnaires ou des partenaires privés, donc on s'intéresse donc vraiment à la bonne cohérence des démarches en phase de construction et exploitation. Cher Cher collègue, avis de la commission sur cet oui, Mᵐᵉ la présidente. Sénateur Jacquin, je salue l'attention portée par les signataires, et, notamment vous, de l'amendement à la sûreté des transports publics, qui est en effet un sujet majeur préoccupation nos concitoyens nous avons d'ailleurs adopté un amendement sur ce point essentiel pour autant cette préoccupation pour majeure qu'elle soit ne me semble pas pleinement avoir sa prévue à l'article trois qui porte sur les modalités de réalisation et de remise des ouvrages construits par la G P. S N C F réseau et S N C F, car les connexions de même les enjeux de sécurité de l'exploitation et la définition d'une trajectoire économique et financière projetée par l'exploitation des Serbes relèvent plutôt de la convention conclue entre les maîtres d'ouvrage et les financeurs prévus à l'article un. Le texte de la Commission comprend bien ces mentions, il faut donc éviter tout doublant qui serait source de confusion. avis défavorable monsieur le rapporteur avis du gouvernement

communs et l'article quarante c'est celui qui consacre un dispositif de vérification donc il me semble que les choses sont satisfaites par la réglementation, la législation actuelle et je vous en demanderai donc euh le retrait. à défaut, j'exprimerai aussi un avis euh défavorable, merci M. le ministre.

Uziel. Mᵐᵉ la Présidente, M. le Ministre, chers collègues, je voulais simplement réagir aux proposs de M. le ministre tout à l'heure, sur les financements apportés par l'état et par les régions dans le cadre des P E R. R. confirme que la majorité régionale pour la Bretagne a eu l'occasion de voter sans doute l'un des 1ᵉʳˢ P E r volets mobilités. On s'est battu pour obtenir une hausse sensible des crédits mais pour autant au regard de l'ordre de grandeur des dépenses en matière de mobilité je pense que là tous les collègues en sont conscients on voit bien que les besoins sont toujours plus importants pour information sur la région bretagne la participation de l'état s'élève pour la période deux mille vingt trois

ces efforts doivent être toujours amplifiés et au demeurant les ressources fiscales des collectivités et en et en particulier des régions qui sont chefs de file vous les connaissez bien ce sont des recettes assises sur les énergies fossiles qu'il s'agisse de l'ex ou des cartes grises donc là évidemment il y a une aberration à non sens c'est à dire qu'une région très volontaire sur le sujet des mobilités décarbonées je crois qu'elles le sont toutes évidemment va voir ces recettes diminuer très sensiblement pour la région bretagne sur les cartes grises en deux mille en deux mille et donc oui l'état a sans doute raison vous êtes dans votre rôle d'appeler les régions à faire toujours plus mais encore faut il nous en donner les moyens encore faut il en donner les moyens aux collectivités c'est le sujet de l'autonomie fiscale et financière on pourra y revenir lors du l f mais c'est le sujet je me permets d'y revenir du versement de mobilité additionnelle, qui constitue l'une des solutions attendues par les régions dans leur diversité et dans le respect de leur sensibilité politique, Donc j'espère que vous aurez l'occasion de nous apporter des éclairages sur ce sujet. Je vous remercie. Cher collègue, nous allons, M. le Ministre, je vous en prie. Je peux pas être trop long sur ce sujet qui va, mais bien sûr, euh et c'est d'ailleurs des articles suivants ou des amendements suivants, notamment de la conférence de financement que le Sénat et la Commission a souhaité ajouter. J'aurais pas forcément formulé les choses ainsi, mais je comprends la demande qu'il y ait une visibilité. On a parlé tout à l'heure sur les questions d'investissement, mais c'est parfaitement légitime, même si cet investissement, je doit être évidemment conjoint, donc c'est tout à fait normal, demander à l'état ce qui est prêt à mettre sur la table, il faut demander à l'ensemble des collectivités, est ce qu'elles sont prêtes à mettre sur la table, et ça n'est pas polémique, c'est un fait et il faut qu'on se pose aussi la question parce que soyons honnête, c'est ce qui a manqué dans euh la préparation du Grand Paris Express comment on financera l'exploitation à mesure que cette offre de transport puisque c'est là le but et c'est ça le souhait partagé augmentera je n'ai aucun tabou sur ces sujets nous aurons l'occasion d'en discuter au moment du projet de loi de finances et j'ai eu l'occasion de dire C'est sur ce point que je voulais m'étendre 1 s que je voulais m'étendre 1 s lors du congrès des régions France où j'étais dans votre belle région à Saint Malo, il y a quelques semaines que j'étais prêt et même disponible rapidement pour ouvrir cette question des financements

chers collègues cet amendement fait directement suite à nos échanges à l'instant monsieur le ministre donc je ne doute pas que vous émettez dans ces conditions un avis favorable il s'agit de garantir un plan de financement pour les termes qui verront le jour un plan de financement complet et sur la partie, évidemment, investissement nous en sommes tous et tous d'accords les infrastructures mais également sur la partie fonctionnement exploitation parce que c'est souvent l'angle mort. on On a eu l'occasion d'en discuter très longuement. en commission et je tiens ici à saluer une nouvelle fois l'initiative du rapporteur. pour la mise en place de cette conférence de financement parce que, comme nous sommes très largement contraints par l'article 40, il faut être imaginatifs et créatifs donc notre collègue Tabar Tabar a a a su trouver cette bonne idée ce bon véhicule qui nous autorise justement ces débats de fond qui sont absolument indispensables, si on veut traduire dans les faits nos ambitions politiques en faveur du développement des mobilités décarbonées donc là ce rapport fait partie des briques que nous appelons de nos vœux pour donner de la lisibilité et de la lisibilité aux acteurs sur les financements nécessaires je vous remercie sept madame la présidente monsieur le sénateur zn a malgré les paroles très agréables que vous avez eues à mon égard et et je vous remercie Euh, je ne

des E M. aussi bien dans les investissements mais bien sûr et surtout dans dans les dépenses liées à leur exploitation dans le futur c'est bien pour cette raison que j'ai proposé cette commission et vous l'avez rappelé à la Commission de prévoir l'organisation de cette conférence. il ne semble pas opportun de prévoir avant même qu'il ait commencé. et à quoi elle aboutit, c'est à dire qu'il n'est pas réaliste de demander au gouvernement de prévoir, à l'issue d'une conférence qui aura lieu dans huit mois, tout au pluss, un plan de financement complet pour chaque Er M, alors que leur périmètre n'a pas été encore arrêté. Les besoins nouveaux n'ont pas été encore pleinement estimés par les collectivités territoriales compétentes, ce plan de financement devra en outre faire l'objet de discussions entre les acteurs locaux. Donc, je pense que c'est un petit peu prématuré pour autant, nous conservons le même objectif et la même volonté. Merci M. le rapporteur, M. le ministre. Oui, Mᵐᵉ la Présidente, je pas sûr que le gouvernement aurait été, si la procédure avait été autre initiative de cette idée de conférence j'en accepte l'augure c'est maintenant dans le texte issu de la commission Euh conférences et rapports je pense que ça fait beaucoup et que ça s'emboîte difficilement et que les briques accumulées comme vous l'avez dit, et pour reprendre votre expression, commencent à faire un mur relativement épais.

raison que M. le Ra rapporteur. Sur le fond, je veux pas qu'on contraigne trop le calendrier ou qu'on l'enferme dans une sorte de modalité unique parce que encore une fois et ce n'est pas une façon de ne pas traiter le sujet, il faudra que chaque terme, c'est l'essence et c'est la lettre d'ailleurs comme l'esprit de la loi chaque terme devra faire l'objet d'un plan de financement et d'un plan d'investissement par les collectivités qui le portent et d'une validation par l'état, en l'occurrence par la ministre chargé des transports, il est évident que les collectivités vous l'avez tous dit nee soumettrons pas à la validation du gouvernement, un plan d'investissement et un plan de financement qui seraient incomplets et sans savoir ce que l'état mettrait ou ce que Les ressources qui pourraient être dégagées apporteront comme financement à ce service express régional métropolitain en investissement en exploitation. Donc je pense que, de toute façon, la nature même du processus fera que la question du financement sera abordée discutée et réglée avant la validation de chaque je ne suis pas pour l'alourdissement des outils en ce sens. vous l'aurez compris, donc je vous demanderai le retrait pour cet amendement à défaut, J'émettrai également un avis défavorable Prenons bonne note des engagements de monsieur le ministre sur le sujet également des proposs du rapporteur et dans ces conditions nous retirons l'amendement

madame la présidente monsieur le ministre chers collègues on a eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises le sujet des moyens gestionnaire d'infrastructures en l'occurrence s n c f réseau est au cœur du fait de nos débats même si dans le cadre de ce véhicule législatif nous ne pouvons pas entrer dans les détails financiers on a eut l'occasion de le dire en évoquant le rapport particulièrement alarmant de l'autorité de régulation des transports de juillet deux mille vingt trois donc encore une fois ce n'est pas un document ancien sur les besoins financiers en matière de régénération de modernisation du réseau et parce que c'est l'objet de la présente proposition de loi des investissements nécessairement massifs dans les années qui viennent pour le développement des ermes dans ces conditions il nous semble absolument indispensable dans la foulée de débats quii ont eu lieu d'ailleurs sur le mandat précédent de réviser le contrat de performance qui lie S, N, c c f réseau et et l'état et de réviser et de s'attaquer au carcan que constitue la règle d'or c'est l'objet de cet amendement en l'occurrence nous nous pensons as que le plafond du ratio d'endettement devrait être révisé à la hausse de s

pour le secteur des transports moins vingt huit pour cent nous en sommes évidemment très loin et le développement du ferroviaire nous permettra d'atteindre ces ces objectifs à condition d'y mettre les moyens et c'est l'objet de cet amendement cher collègue monsieur le rapporteur il y a un sous amendement que je vous demande de présenter c'est C'est bien cela, Mᵐᵉ la Présidente, il y a un sous amendement qui précise, comme le suggèrent les auteurs de l'amendement, le rôle de la conférence nationale de financement proposée par l'article trois inséré en commission dans le processus de révision du contrat de performance entre N C F réseau et l'état il supprime par ailleurs la mention relative règle d'or qui s'applique à la S N C F réseau la conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains comme son nom l'indique d'ailleurs a vocation à trouver financement des E R Ms les plus adaptés et non pluss largement à revoir le modèle économique et financier du groupe N C F qui dépasse largement son périmètre. de réflexion et comme j'imagine, Mᵐᵉ la Présidente, que votre prochaine question est de connaître mon avis sur l'amendement, je vous proposee un avis favorable sous réserve de l'adoption du sous amendement 60.

le plus problématique vu du gouvernement de l'amendement proposé par m jacquin défendu par m usn a je suis défavorable à l'ensemble parce que bien sûr nous partageons la préoccupation du réinvestissement de travailler sur le contrat de performance qui doit être je je le crois je l'ai dit tout à l'heure actualisé évidemment j'en rendrai compte au Parlement, au Sénat comme à l'assemblée nationale je crois que c'est un objet quii est évidemment connecté au Er mais qui est beaucoup plus large quand bien même nous ne discuterions pas de cette proposition de loi nous aurions besoin de réinvestir notre réseau et de définir une trajectoire pluriannuelle comme l'a indiqué la 1ʳᵉ ministre, avant même que cette proposition de loi issue de l'assemblée existe donc je ne voudrais pas qu'on confonde en quelque sorte les deux sujets et qu'on lit le travail sur le réseau qui est indispensable, et le réinvestissement sur le réseau est nécessaire avec la question des services express régionaux métropolitain, c'est la raison pour laquelle pour laquelle je suis défavorable à l'amendement et par conséquent au sous amendement, même s'il atténuerait un petit peu la difficulté. M. le rapporteur. Merci M. le ministre, M. Zadeh Ation, de vote. Bah, vous l'aurez compris, M. le ministre, et je pense que c'est très largement partagé sur ces bancs. Euh, soucieux de l'équité territoriale de garantir un aménagement équilibré de nos territoires, nous sur les dessertes ferroviaires. Euh, nous voulons tenir les deux bouts de la chaîne à la fois sur la régénération, la modernisation du réseau et sur le développement des Ser Mes qui vont constituer un service à valeur ajoutée pour nos concitoyennes et nos concitoyens, donc, évidemment, nous nous voulons faire le lien entre ces deux sujets. Ns sommes évidemment favorables au sous amendement de M. le rapporteur et nous le remercions pour cette initiative

la concertation il est prévu qu'en cas de modification du schéma d'ensemble du réseau de transport grand paris doivent être recueillis doivent être recueillis un certain nombres d'avis dont celui du syndicat mixte Paris Métropole et de l'atelier international du Grand Paris qui n'existe plus ni l'un ni l'autre, donc il s'agit l'un ni l'autre, donc il qu'il faut entendre. plus globalement et pluss De façon plus importante, sur cet amendement, je voudrais parler du périmètre géographique de consultation puisque, à l'origine de la loi du Grand Paris, il s'agissait de faire une consultation sur la globalité du schéma et donc sur la totalité des Franciliens et la totalité de l'île de France aujourd'hui, l'ensemble des lignes sont soit commencées soit en travaux, soit presque terminés, il s'agit juste de modifications et donc je suggère dans cet amendement que On revienne en fait au droit commun pour les modifications du schéma et que en plus de l'association des maires d'île de france et d'île de france mobilité seules les collectivités territoriales et les p c i dont le territoire est impacté soient consultés ce qui permett plus de facilité et d'agilité merci madame la présidente à l'avis de la commission sur l'amendement madame la présidente mesdames les présidentes sur le l'amendement cinquante six il actualise opportunément les modalités de consultation en cas de modification du schéma d'ensemble du réseau de transport du grand paris donc il allège le processus initial qui n'a pas lieu d'être compte tenu du stade d'avancement du projet donc il n'y a aucune raison pour ne pas donner un avis favorable monsieur le rapporteur avis du gouvernement sur le madame la présidente je ne voudrais pas qu'on fasse croire qu'il y a une modification qui est envisagée dans les prochaines semaines dans les prochains mois j'avais une petite réticence sur cet amendement à ce titre néanmoins s'il devait y avoir une modification les modifications que vous proposez sont assez pertinentes et de bon sens donc j'émettrais un avis de sagesse sur cet amendement madame la présidente bienveillant merci votre sagesse merci votre sagesse est toujours apparemment bienveillante monsieur le ministre merci beaucoup je vais mettre aux voix l'amendement cinquante six avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement d'un

donne un délai de 10 ans pour réaliser les enquêtes publiques des des D U P Euh. Or, il n'est pas permis de définir avec certitude si ce délai de 10 ans pour réaliser les enquêtes court à compter du délai d'approbation initial du schéma d'ensemble ou à compter des décrets approuvant des modifications de ce schéma d'ensemble, donc pour lever cette incertitude je vous propose cet amendement il serait opportun d'ajouter expressément le terme modification à l'article quatre de la loi sur le Grand Paris afin d'éviter toute incertitude et de consolider juridiquement les procédures Mᵐᵉ la Présidente, M. le rapporteur, votre avis, oui, Mᵐᵉ la Présidente, je vais donner un avis favorable puisque cett amendement permet de lever une ambiguïté et c'est bien de lever les ambiguïtés.

pour qu'ils fassent l'objet d'une prise en compte spécifique à travers le forfait national le groupe écologiste s'oppose donc à toute nouvelle tentative de contournement de cette loi qui remettrait en cause l'objectif de réduction de cinquante de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers fixés pour deux mille trente et un les projets de serm quand ils réalisent des infrastructures nouvelles n'ont pas à être exonérés de la trajectoire du il participe bien le cas échéant au recul des terres agricoles et des espaces naturels mais bien sûr ils ne doivent pas non plus impacter directement l'enveloppe des communes d'implantation afin d'éviter la double peine pour les territoires qui seraient privées d'une très grande part de leur capacité à agir en à cause du poids des infrastructures. c'est pourquoi ces projets doivent être recensés au sein des enveloppes régionales dans le cadre du forfait régional car les Er Ms ne se traduisent pas forcément par la création de

merci cher collègue un amendement identique présenté par monsieur jacquin l'amendement vingt cinq vient d'être parfaitement défendue par m erni merci beaucoup chers collègues avis de la commission sur ces deux amendements identiques

Cette option présente deux principaux avantages premièrement, la section des travaux publics du Conseil d'état pourra se prononcer en formation consultative sur l'utilité publique du projet. projet. Deuxièmement, en cass de recours il n'y a plus qu'un seul degré de juridiction compétent le Conseil d'état et non pas trois comme c'est le cas pour les arrêtés préfectoraux, l'urgence écologique et le des F-des F m par c'est l'habitude, exige en effet une réponse rapide. Cette disposition peut faire économiser plusieurs années de contentieux Cette disposition permett aussi aux projets de E R M d'être considérés comme des projets d'envergure nationale ou européenen dans le cadre des règles encadrant le zéro artificialisés nette pour lever tout malentendu sur cette question. je tiens à mentionner deux éléments d'une part cette comptabilisation dans l'enveloppe nationale est une simple possibilité qui n'a pas vocation à être systématique et d'autre part le volume global de cette enveloppe qui est de douze mille cinq cents hectares n'augmente pas on réfléchit donc toujours à niveau d l'artificialisation constante j'espère que les choses que les choses sont claires maintenant et que c'est uniquement dans un souci de rapidité pour ne pas retarder un certain nombre de projets qu'on a souhaité. apporter ces modifications au texte initial. Donc, je vous donne un avis favorable, mais je suis sûr que, avec les explications précises que j'ai pu vous donner, bien sûr défavorable, vous allez retirer vos amendements, en tout cas je le souhaite fortement.

euh du coup me fait donner un avis favorable à ces amendements pourquoi parce que sur les l'obligation de déclaration d'utilité publique par la procédure Conseil d'etat, c'est vrai, M. le rapporteur, que ça a un avantage et que ça a réduit les délais de contentieux et les niveaux de recours ce que je partage, je ne sais pas, c'est le but qui était poursuivi et ce que je partage en revanche, la procédure elle même de passage en Conseil d'état est plus longue que celle de l'arrêté préfectoral au nom du gouvernement, qu'on garde la possibilité d'avoir des procédures qui passent aussi par arrêté préfectoral et qu'on ne soumette pas l'ensemble des procédures serm par avance au niveau de la D U P. après passage après avis du Conseil d'etat, pardon et par décret en Conseil d'état c'est la raison pour laquelle je voyais peut être pas exactement les mêmes motivations, mais un avantage à soutenir ces amendements euh manifestement il y aura encore un peu de travail pour partager les objectifs, un avis favorable du Gouvernement, qui

l'assemblée la présidente l'assemblée a intégré une demande de rapport assez opportun sur la réouverture de la compétence là je viens plaider pour des territoires oubliés de la lomme qui sont certains espaces peu denses dans lesquelles les ressources en versement mobilité sont très faibles par exemple, sur mon ancienne intercommunalité de 50 communes 20 habitants lorsqu'on lève le versement mobilité on ne peut pas récolter plus de 100 € de ressources fiscales, impossible de mettre en œuvres des politiques de mobilité. donc je voudrais en profiter pour à cet endroit req questionner notre hémicycle sur certains territoires qui sont en difficulté pour mettre en place des politiques de mobilité mille vingt et un consacré aux mobilités dans les espaces peu denses je souligner que la sortie d'un modèle de mobilité centré presque exclusivement sur la possession et l'utilisation de la voiture individuelle étaient possibles dans ces espaces bien que de nombreux obstacles restent à surmonter et au premier rang le manque de moyens financiers Je rappelle que la Lom a donné la faculté aux communautés de communes institué le V. M. M, mais que cette contribution, comme je l'ai dit, est très inégale en fonction des activités et des emplois. que l'on trouve sur ces territoires, il est donc important de consolider ces données sur les P. C I. en capacité ou non, de levée du versement mobilité et de trouver des solutions pour ce ne pouvant ne pas disposer de cette ressource L'idée d'une fraction de I C P. E qui serait dévolue à ces territoires pourraient constituer une solution pour financer des services de mobilité dans ces territoires ruraux tout en permettant de donner une vraie finalité environnementale à cette taxe acquittée par les automobilistes. la raison pour laquelle nous demandons que le rapport prévu à cet article soit simplement étendu au soutien que le Gouvernement compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses. Ce rapport étudiera en particulier la possibilité de financer les services de mobilité. Cher collègue, je vais demander l'avis de la commission. Sénateur Jacquin. Et puis je, si on donne un avis favorable, c'est qu'on veut être en cohérence avec la demande de rapport que nous avions faite euh au moment du climat résilients Sr, ce même sujet D'ailleurs, j'aimerais savoir où en est ce rapport, Moi j'ai pas eu connaissance Moi, je de sa publication. Donc, si jamais M. le ministre de l'information, ça pourrait nous intéresser en tout cas pourrait être cohérents par rapport à ce que nous avons voté et donc demandé dans le climat et résilience euh je propose de donner un avis favorable à la demande du sénateur

Merci M. le ministre, M. Jacquin, pour une explication Je serais ravie que le rapport demandé dans la loi climat résilience sorte effectivement dans quelques semaines, mais un tiens vaut à vaut mieux que deux tu l'auras, je préfère maintenir cet amendement. Nous sommes en passe d'obtenir enfin ce document attendu depuis plusieurs années. Merci, vous cher On va l'avoir et on va l'obtenir très prochainement mais je pense que c'est C'est vraiment et particulièrement utile à la fois d'évaluer sur ces zones Pede effectivement, la question du versement mobilité et, en tout cas, du financement de ces de ces zones, de ces zones peu dense et aussi sur le bilan de la prise de compétences. compétences. que c'est particulièrement intéressant qu'on puisse avoir ce bilan de la prise de compétences. On sait aussi qu'il y a eu une action d'un certain nombre de régions, parfois pour bloquer cette prise de compétences au niveau des Oem et donc de voir aussi l'opportunité de réouvrir et cette possibilité de prise de compétence par des m peut se poser je pense don que ce rapport ou ces rapports du coup s'il y en a s'il sihon particulièrement importants monsieur le président gontard je mets aux voix cet amendement cinquante et un qui a reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement qui vote pour